La séance est reprise J'informe le Sénat une candidature en remplacement d'un membre démissionnaire pour siéger au sein de la CMP chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique a été publié cette candidature sera ratifié si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue de notre règlement, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à faire évoluer la gouvernance de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à créer les instituts régionaux de formation présentée par Madame Sabban, Samantha Cazebonne la procédure accélérée a été engagée sur ce texte dans la discussion générale, la parole est à Madame Samantha Cazebonne, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Garde l'immense Très bien monsieur le président merci. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, j'aimerais commencer par tous vous remercier monsieur le ministre, monsieur le rapporteur également chers collègues représentants des Français établis hors de France pour votre engagement et votre soutien. Et ce n'est pas seulement en tant que sénatrice que je vous adresse mes remerciements, mais également en tant qu'ancienne proviseur des lycées français au Maroc et en Espagne. Si nous avons parfois dans cet hémicycle des points de vue divergents qui font la richesse d'un débat parlementaire passionné, une synagogue, une citation de Nelson Mandela, sur laquelle nous pouvons nous retrouver unanimement l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, la France depuis maintenant des décennies, a fait de l'enseignement français à l'étranger, un outil d'influence et de rayonnement de notre pays. Nous, Français de l'étranger sommes particulièrement fiers que dans 138 pays la France puisse porter ses valeurs, son histoire, son savoir-faire éducatif et pédagogique, ainsi que la francophonie. Si notre réseau d'enseignement scolaire à l'étranger, défend la place de la France à l'international, il s'est également s'enrichir du multiculturalisme du plurilinguisme de l'inclusion du respect de la différence de l'égalité entre les femmes et les hommes en y forge des esprits critiques on y défend des convictions humanistes et des savoirs qui confère à nos élèves une richesse intellectuelle rechercher dans les plus grandes écoles et universités internationales. Il suscite l'intérêt bien au-delà des familles françaises sur tous les continents, des familles qui recherchent et rejoigne notre réseau scolaire français et c'est 552 établissements homologués dans le monde. Les parents d'élèves sont de plus en plus nombreux à vouloir rejoint notre réseau à vouloir dans leur pays une école française à cette attente, nous devons répondre présent augmenter notre offre scolaire française afin de se positionner comme alternative crédible au modèle anglo-saxon chinois, turcs, qui se développe de manière exponentielle, c'est porté par cette belle et noble ambition que permettent, pardon, de permettre à toujours plus d'enfants français à l'étranger d'avoir accès à travers le monde à un enseignement francophone plurilingue ouvert sur les cultures des pays d'accueil, que le président de la République s'est engagé à doubler les effectifs de ce réseau dans son discours sur la francophonie, du 20 mars 2018. Ce réseau est une chance pour la France et son influence, vous seriez d'ailleurs surpris du nombre de personnalités du monde de la culture, des arts, des sciences de l'entreprise, de la politique, qui ont reçu une éducation au sein de nos écoles françaises à l'étranger, ce sont des milliers d'anciens élèves de toutes nationalités établis partout dans le monde et qui, grâce à cette éducation cet attachement à la France crée des relations économiques, artistiques diplomatiques, politiques avec la France et leur pays d'origine, monsieur le ministre, je vous c'est totalement convaincu par cette ambition du président de la République, vous qui l'a porté au quotidien sur le terrain depuis 5 ans déjà, et si vous me le permettez, en tant qu'ancien élève de ce réseau, vous le connaissez certainement mieux que quiconque. Nous devons donc nous fixer des objectifs ambitieux : gagner en compétitivité et en puissance et c'est pour cela qu'aujourd'hui cette PPL se met au service de ce réseau et de son développement, tous les gouvernements en place ont assumé de mener ces 15 dernières années une politique qui permettait aux établissements au statut des partenaires de se développer. C'est non seulement un faux procès, mais un procès mensongers ou en méconnaissance que de dire que ce gouvernement tiendrait tendrait pardon à privatiser ce réseau scolaire, il suffit de reprendre les rapports d'ancien sénateur des Français de l'étranger : je pense à André Ferrand, qui a beaucoup oeuvré pour ce réseau, mais également à Claudine Lepage au rapport de la Cour des comptes des inspections générales de l'éducation nationale et des Affaires étrangères, ou bien encore celui des sénateurs, Rémi Féraud et Vincent Delahaye, en 2018 pour vérifier que, depuis près de 15 ans, ce sont ces établissements partenaires homologué par l'Éducation nationale et encadré par le MAE qui ont fait croître le plus : les effectifs des élèves des personnels titulaires de l'Éducation nationale en détachement ou d'enseignants locaux. La volonté, à l'époque n'a jamais été de soutenir le développement, pour répondre à la demande de croissante des familles mais de maintenir l'existant tout en augmentant de 2008 à 2016 de 60 % les frais de scolarité pour les familles, et ce n'est pas moi qui le dit, mais les chiffres de la Cour des comptes Le rapport Lepage Corderie en 2014 qui mettait en avant le constat édifiant : jamais les frais de scolarité n'avait autant augmenté. Lui, ce gouvernement il a augmenté, mais la subvention publique à hauteur de 150000 euros, c'est inédit, une hausse. Cette hausse pardon a fait passer de 500 millions à 650 millions l'aide accordée aux élèves, aux familles, aux personnels, tous statuts confondus et aux établissements, cela a permis d'éviter des départs d'enfants scolarisés depuis des années dans nos et dans leurs établissements, des licenciements et des fermetures oui soyons fiers que pour la première fois sous cette majorité l'ensemble et je dis bien l'ensemble des familles et donc des élèves de ce réseau, qui en ont fait la demande et pu être aidé des familles françaises ont été soutenues avec plus de 50 millions d'euros supplémentaires, tout comme les familles étrangères aidées à hauteur de 50 millions d'euros qui ont permis de soutenir nos établissements. Mais au-delà du soutien financier dans le cas du développement voulue par le président, il nous a, il nous faut désormais prendre à bras-le-corps la dimension qualitative de ce réseau développé oui mais développer bien et avec des compétences professionnelles certifiées grâce à des formations qualifiantes qualifiantes ou diplômantes après ces quelques points de contexte j'en viens désormais à la PPL qui nous réunit aujourd'hui et qui vise à faire évoluer la gouvernance des missions et l'émission, pardon de l'AFE est à prévoir une base juridique pour la création des instituts régionaux de formation, l'article 1er de la PrEP, elle vise à prévoir la participation au conseil d'administration de la greffe en qualité d'expert, d'un représentant des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger et d'un représentant des associations flammes les anciens élèves qui représentent grâce à l'Union, elle FM 148 associations locales pourront siéger en qualité d'expert et apporter leur éclairage, donner leur avis et faire des propositions pour les réseaux, il me semblait indispensable que nous puissions partager de manière régulière,

Les flammes, fleuron de l'enseignement français et des valeurs françaises avec nos alliances et nos instituts français doivent trouver un nouveau canal d'expression pour faire entendre leurs enfants, leurs attentes, leurs besoins et partager leur savoir-faire exceptionnel qui réunit aujourd'hui près de 14000 élèves dans 173 associations implantées dans 39 pays, l'article 2 vise lui a modifié la proposition des représentants de chaque catégorie pour rehausser la part de la représentation des parents d'élèves et prévoir expressément une représentation des parents gestionnaire, parce que notre réseau ne serait rien sans ses acteurs il est, il en est, pardon, qui aujourd'hui ne sont pas reconnus à la hauteur de leur engagement, il me paraissait indispensable qu'à travers ce texte nous remettions un peu d'équité dans la représentation des acteurs essentiels sans ôter de légitimité à ce dans ce réseau. sans lesquelles nous pourrions un fonctionner, c'est-à-dire les enseignants et leur représentation syndicale. Sur cette partie je vous proposerai d'ailleurs un sous-amendement afin que les représentants des parents d'élèves les plus représentatifs, voient leurs droits et pouvoir d'expression renforcée. Enfin, les articles 3 et 4 visent à étendre les compétences de la EFE et à modifier le code de l'éducation pour prévoir la gestion par l'opérateur public des instituts régionaux de formation. Les 16 instituts régionaux de formation attendu est déjà en état de fonctionnement n'attendent que nous parlementaires pour prendre enfin leur élan et faire de ce réseau, un réseau qui sera assurée dans un proche avenir des formations initiales et continues identique à celle dispensée en France, les enseignants qui sont nombreux chaque année à rejoindre ce réseau sont des acteurs essentiels ainsi que leurs collègues, personnels d'encadrement, d'éducation et administratifs je tiens évidemment à les saluer et les remercier pour leur travail, et particulièrement pendant 7 ans de crise sanitaire parce que les familles sont également de plus en plus exigeantes, compare les modèles d'éducation pour aller vers ceux qui auront, qui seront démontrer le meilleur pour leurs enfants, il nous faut permettre à nos enseignants, de gagner en compétences en expérience en méthode innovante la EFE aura pour mission de faire vivre et prospérer IRF des instituts régionaux de formation, l'agence devra coordonner sa propre ingénieur et de formation avec celle proposée par d'autres opérateurs, tels que la Mission laïque française et la Fleck ou des établissements conventionnés comme à Mexico partenaires comme Turin comme à Tunis par ces instituts devront à terme Jean nourrit l'espoir et je le soutiendrai permettre au personnel titulaires de l'Éducation nationale ou stagiaires de valider leurs acquis d'expérience de réaliser leur stage de titularisation et de faire reconnaître des qualifications sans avoir à rentrer en France, ce qui jusqu'alors ouvrez le risque de perdre son poste à l'étranger, les attentes sont fortes et les enjeux sont d'importance, chers collègues, l'enseignement français à l'étranger, attend les familles attendent les personnels attendent mais surtout et avant tout les élèves nous attendent alors Dondo toutes ses chances à ce réseau de conclure à compter parmi les meilleurs au monde et se développer pour permettre à davantage d'élèves d'en bénéficier et à la France de rayonner en déployant la plus belle des diplomatie d'influence notre modèle d'éducation français merci, cher collègue. Non, non, monsieur le ministre, c'est pas vous qui décidez, merci madame, merci chers collègue, je le dis tout de suite pour la suite des débats, 2 minutes c'est 2 minutes c'est pas 2 minutes 30 ni 2 minutes 40, d'autant qu'il y a un texte derrière vous, encore. Allez, la parole est à monsieur Bruno Sido, rapporteur de la commission des Affaires étrangères de la Défense des forces armées pour 10 minutes. Quelle que soit la volonté du ministre dix minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Cette proposition de loi dont notre collègue et Samantha Cazebonne vient de présenter les objectifs procèdent aux ajustements nécessaires pour permettre à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, d'accompagner la croissance de son réseau dans l'objectif de doubler les effectifs à l'horizon 2030, le réseau de l'enseignement français à l'étranger et le fleuron de notre diplomatie culturelle et d'influence, comme vient de le dire, ma collègue, c'est un réseau qui permet d'abord aux enfants français expatriés de disposer d'une éducation de qualité à l'étranger et de conserver un lien fort avec la France, c'est aussi un réseau mondialement reconnu comme dispensant un enseignement d'excellence, un réseau dont le pouvoir de rayonnement et sans équivalent qui fait la fierté de notre pays, ce réseau démontre en effet sur les 5 continents et dans les 138 pays où il est implanté que nous sommes encore une nation dont la langue et la culture sont omniprésentes dans le monde, les anciens élèves, dont le nombre est évalué à 600000 dont de nombreuses personnalités françaises et étrangères sont autant d'ambassadeurs à la, à, vis de la langue de la culture et des valeurs de la France en 30 ans les effectifs du réseau ont plus que doublé, passant de 165000 élèves en 1990 à 375000 aujourd'hui, l'ambition du président de la République et de doubler à nouveau les effectifs, c'est-à-dire d'accueillir 700000 élèves d'ici 2030, on ne peut qu'approuver cet objectif ambitieux qui contribue à ce que le soft power est ainsi un nom en français, le pouvoir d'influence ou le pouvoir de convaincre dont on voit aujourd'hui qu'il est au coeur de la compétition, voire de la confrontation entre puissances, l'éducation est aussi un combat pour les valeurs très concurrentiel c'est évident dans l'enseignement supérieur mais c'est aussi le cas au niveau des écoles, des lycées, on connaît la force des réseaux anglo-saxon et l'activisme de la Chine, la multipolarisation du monde démultiplient le nombre d'acteurs en compétition dans un Champ qui doit être considéré comme une composante à part entière de notre diplomatie, au-delà des effets d'annonce, toutefois, quels sont les moyens réellement mis en oeuvre pour consolider et développer le réseau de l'enseignement français à l'étranger, l'État a investi au total 520 millions d'euros de crédits budgétaires annuels dans cet enseignement, la commission des Affaires étrangères et de la défense dénonce régulièrement dans ses travaux, les limites de la stratégie suivie en l'absence de croissance suffisante des moyens budgétaires nous nous étonnons également de la stagnation de la non-qu'on peut se consommation de l'enveloppe des aides à la scolarité dans un contexte d'augmentation des effectifs par ailleurs entre 2016 et 2021 le nombre d'enseignants a baissé de 21 % pour les personnels expatriés et de 7 % pour les personnels sous le statut de résident le ministère de l'Éducation nationale promet 1000 détachements supplémentaires avant 2030, mais ce chiffre, même s'il est atteint, sera loin d'être suffisant pour accompagner la croissance du réseau, un verrou important réside dans l'interdiction faite à la EFE d'emprunter à moyen et long terme, cette interdiction n'a toujours pas exister à sa création en 1990 l'AFE étaient autorisés à emprunter ce qu'elle a pu faire jusqu'en 2011 étant classé comme organismes divers d'administration centrale, les fameuses elle a été ensuite été privé de cette capacité au nom de la lutte contre l'endettement public, or le développement du réseau doit passer par une croissance non seulement des établissements partenaires mais aussi des établissements en gestion directe, qui sont le coeur du dispositif et ont besoin de réaliser d'opérations immobilières par ailleurs pour les établissements conventionnés et partenaires, le nouveau dispositif de garantie de l'État est moins favorable que celui qui préexistait à travers à travers de l'association nationale des écoles françaises à l'étranger, la tout ceci est en contradiction avec les ambitions de développement du réseau dans ce domaine, le Parlement était s'empêcher d'agir par l'article 40 de la Constitution, mais nos débats permettront peut-être d'obtenir des éclaircissements, Monsieur le Ministre, car des avancées sont nécessaires, l'agence ne peut recourir qu'aux avances de France Trésor et encore à titre exceptionnel dans l'attente de la mise en place d'un nouveau mécanisme de financement, un groupe de travail chargé de réfléchir à ce niveau, mais nouveau mécanisme qui pourrait nous dit-on être fondé sur une mutualisation entre établissements, mais comment imaginer puiser dans les réserves d'un établissement issu des écologistes pour financer les travaux de dans d'autres établissements, les familles qui financent 64 % du fonctionnement des oeufs GD le comprendraient mal l'interdiction du recours à l'emprunt, et d'ailleurs d'autant plus contestable qu'elle intervient dans le contexte d'un financement majoritaire par les familles l'AFE n'étant pas comme les autres Hodac des organismes divers d'administration centrale financée majoritairement par l'État dans ce contexte, les avancées permises par la proposition de loi de notre collègue, Samantha Cazebonne sont bienvenues, il s'agit tout d'abord d'élargir la gouvernance de l'agence, en y associant davantage les parents d'élèves, cette évolution est légitime : je viens d'évoquer le rôle prépondérant des familles dans le financement des eaux GD dans l'ensemble du réseau, ce sont 81 % des coûts de fonctionnement qui sont financées par les familles, la proposition de loi permettra à 2 représentants de parents d'élèves supplémentaires de siéger au conseil d'administration et pour respecter les grands équilibres fixés par la loi, le nombre de représentants de l'État augmente également, ce qui portera le nombre d'administrateurs de la EFE de 28 à 31 ce n'est pas un bouleversement, mais un ajustement bienvenu je vous proposerais simplement un amendement mettant l'accent sur la notion de représentativité des fédérations de parents d'élèves, la proposition de loi étant par ailleurs la participation au conseil d'administration à 2 des membres, sans voix délibérative, un représentant des associations d'anciens élèves, un représentant des associations de France de français langue maternelle flamme et, à l'initiative de la Commission a représentant de l'association nationale des écoles françaises à l'étranger, la la proposition de loi complète, enfin les missions de la EFE en ouvrant de nouveaux dispositifs de formation, elle met en place des instituts régionaux de formation qui seront gérés directement par l'AUF le développement du réseau homologué nécessite en effet de disposer de personnels qualifiés qui soit garant de la qualité de l'offre d'enseignement, or la plupart des personnes, recruter des personnels recrutés localement, ne sont pas titulaires de l'Éducation nationale, l'enjeu est majeur puisqu'il s'agit de préserver la qualité qui fait la réputation de l'enseignement français à l'étranger, dans le contexte d'un développement accéléré du réseau, les instituts régionaux de formation pourront proposer non seulement la formation continue, mais aussi des cursus diplômant à un public élargi pour clarifier ce Champ d'action, la commission a adopté un amendement tendant à leur donner prioritairement pour objet de former les personnels et futur personnel, elle a également souhaité que ces formations soit un outil de promotion de la francophonie. Mes chers collègues, je vous propose de soutenir ce texte, qui vient conforter la dynamique de l'enseignement français à l'étranger, je suis heureux qu'il nous donne l'occasion de débattre d'un sujet essentiel suivi attentivement par notre commission mais sur lequel les textes législatifs sont rares, or vous l'aurez compris, il s'agit d'une question majeure intéressant environ 3 millions de Français expatriés et dont les dimensions diplomatique et stratégique ne saurait être négligé, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, et merci pour votre concision, ça n'est pas du tout un commentaire par rapport au ministre mais c'est son. Tour Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie à la parole. Bien, monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame la sénatrice Samantha Cazebonne mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices. Jules Verne, Antoine de Saint-Exupéry, Victor Hugo, Mermoz, Jean Monnet Stendhal, Camus, j'en passe, autant de noms familiers de notre histoire littéraire de notre histoire de France, mais surtout autant de noms qui sont inscrits fièrement au fronton des écoles, des collèges, des lycées de cet enseignement français à l'étranger, partout dans le monde, c'est à cela que l'on mesure d'ailleurs son apport, son apport à la fois pour nos compatriotes établis hors de France, qui trouve là matière à pouvoir faire suivre une scolarité dans les mêmes canons que ceux qui sont accessibles, international, et puis en même temps cette capacité aussi à rayonner à faire en sorte que nous puissions partager cette culture, ce savoir cette capacité d'apprendre avec bien d'autres ressortissants et donc nous avons une ambition qui est partagé, je le sais, sur tous les bancs, ici, qui était réaffirmée par le président de la République, c'était en mars 2018, celle de faire resplendir ce trésor national, et donc c'est ainsi qu'à partir de mars 2018 nous sommes attelés à. Préparer un véritable plan d'action pour le développement de l'enseignement français à l'étranger pour mettre en oeuvre à cette feuille de route qui avait été fixée, celle de doubler à l'horizon de 2030, les effectifs des élèves scolarisés dans les établissements français à l'étranger pour bâtir ce plan d'action cette feuille de route donc aujourd'hui la proposition de loi est une traduction législative qui vient parachever justement les démarches mises en oeuvre, hé bien nous avions déjà à l'époque sollicité Samantha Cazebonne pour pouvoir éclairer les décisions et les actions du gouvernement, nous avions aussi concertés naturellement toutes les parties prenantes, les représentants des enseignants des différents personnels, des parents d'élèves naturellement des des anciens élèves, bref de l'ensemble des acteurs et si la crise sanitaire est passée par là, je crois qu'on peut dire que l'enseignement français à l'étranger, il a résisté, il a résisté grâce à un soutien massif de l'État, si je prends juste les aides directes, ce sont 100 millions d'euros qui ont été mobilisés pour les établissements et des familles en difficulté et pour toutes les familles, j'insiste, qu'elles soient françaises ou étrangères et non seulement le réseau, il a tenu bon, mais il n'y a pas eu de mise de clé sous la porte si je puis dire, mais surtout ce réseau, il a continué à se développer, il compte à ce jour, c'était, rappelez et par le rapporteur et par l'auteur de la proposition de loi 552 établissements il y en avait seulement 522 en 2019, on le voit, c'est donc une expansion qui se poursuit et, donc, après des mois difficiles et qui parfois le demeure, parce que naturellement les élèves scolarisés dans l'enseignement français à l'étranger ont été les premiers. De l'ensemble des élèves français à être touché par la pandémie, parce que nos établissements situés en Chine dès le mois de janvier 2020, naturellement, ont été soumis à des contraintes, et bien que nous avons essayé de limiter au maximum ici sur le sol national, il a fallu s'adapter et je veux rendre hommage là aussi à à l'ensemble de la communauté éducative, alors le texte que qui est examiné cet après-midi est essentiel parce que, il porte sur 3 grands enjeux, la formation des personnels, d'une part, la gouvernance de l'agence la UFE et la réaffirmation d'ailleurs du rôle de l'agence comme vraiment un pivot d'opérateurs publics au service du réseau d'enseignement français alors la formation des personnels. Dès les premières concertations qui avait que que j'ai conduite, c'était en 2019, la question de la formation, elle est apparue central pour créer les conditions, et bien d'une croissance du réseau qui soit, qui se fasse en aucun cas au détriment de la qualité des enseignements et développer le réseau attirer de nouvelles familles par une offre éducative de qualité, c'est ça la réputation, et c'est cette réputation, qu'il faut maintenir conforter et bien sûr la demande que nous puissions justement déployés au service des des enseignants, qu'ils soient titulaires de l'Éducation nationale ou pas, hé bien, une hausse de formation qu'elle soit initiale ou continue, qui répondent à leurs besoins et qui est bien permettent voilà deux continuellement monter en compétences adapter les compétences et la création des 16 instituts régionaux de formation les IRF au service des personnels des 552 établissements est une réponse à ce défi et ces ces instituts pour fonctionner doivent être placés en gestion directe de l'AMF, la proposition de loi a trait également à la gouvernance de la greffe et et en particulier ce qui a été dit-elle conforte et même elle renforce la place des parents d'élèves dans le conseil d'administration, c'est un engagement que j'avais pris en octobre 2019 lorsque nous avons présenté ce plan avec Jean-Yves Le Drian, avec Jean-Michel Blanquer, alors c'est vrai que si j'avais écouté tous les tenants du système, il ne fallait pas le faire, mais c'est très bien de l'avoir fait, c'est très bien de l'avoir fait parce que ses parents d'élèves seront représentés, non plus par 2 représentants mais par qui, 4 représentants, nous voulons marquée aussi par la par la même notre reconnaissance envers des familles qui non seulement font confiance à notre modèle éducatif mais le co-finance par des droits des collages et participe activement à la vie de cette communauté éducative. Je salue également l'entrée au conseil d'administration de l'Agence en en qualité d'expert, et bien d'un représentant des anciens élèves, cela a été dit, rappelé par Samantha Cazebonne ceux-ci incarne les valeurs, l'éducation française et leur parcours partout dans le monde est un témoignage de la qualité de l'enseignement reçu, monsieur le président de la Commission pour saluer votre arrivée parmi nous si les experts seront également composer au sein du conseil d'administration d'un représentant des associations flamme, c'est une bonne chose, vous savez je combien nous sommes attachés à ce dispositif qui permet à des enfants français qui n'ont pas la possibilité d'être scolarisés dans le réseau homologué bien de conserver un contact régulier construit avec notre langue avec notre culture et ce réseau est en train de se structurer de façon formidable à travers une fédération internationale et aujourd'hui, on dénombre pas moins de 160 associations dans 38 pays, j'ai eu l'occasion d'aller à leur rencontre au Portugal dernièrement et j'ai vu hé bien puisque le réseau se se mettait en place après le, comment dire, une installation réussie en Espagne, combien cela répondait à des attentes fortes et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai souhaité que nous puissions augmenter significativement le budget dédié au soutien à ces associations qui est porte qui va être multiplié par 3 en cette année 2022 pour passer à un 1000000 d'euros. Alors les évolutions qui sont proposées vont dans le sens justement du renforcement du rôle du conseil d'administration de l'Agence en tant que pilote stratégique en tant qu'instance de dialogue et il faut dire que le rôle de l'agence lui-même aussi est conforté comme ensemblier du du réseau d'enseignement français à l'étranger comme cheville ouvrière de son développement, l'agence se voient confier de nouvelles missions avec notamment son rôle de conseil et d'accompagnement dans la création de nouveaux établissements qui est partie intégrante d'missions qui désormais lui sont eux assignés par le code de l'éducation, les porteurs de projets, qu'il s'agisse d'investisseurs privés ou d'acteurs associatifs peuvent bénéficier de l'expertise de l'agence grâce au service d'appui et de développement du réseau, le SDR et cette activité est en plein développement actuellement une centaine de dossiers de demandes d'homologation, ont été déposées pour la campagne 2021 2022 il y a un tiers sont suivis par le dire et puis la UFE est également partie prenante du nouveau dispositif d'octroi de la garantie de l'État aux emprunts immobiliers des établissements partenaires est conventionné, à ce moment-là, je tiens à saluer l'action qui était conduite par le sénateur Ferrand, qui était de nombreuses années à la tête de la nef et il est vrai qu'il n'était guère possible de pouls de, de, de continuer l'action de la nef, sous la forme qui avait été originellement la sienne, mais nous avons et et ça j'ai j'ai tenu à ce que on puisse préserver néanmoins le savoir-faire qui avait été mis en place au sein de la MNEF et ainsi le fait que la puissent également avoir ce regard d'expert au sein du conseil d'administration, le FE me paraît très précieux puisque la UFE elle-même sera partie prenante du nouveau dispositif d'octroi que j'évoquais et je voulais signaler d'ailleurs que nous allons réunir pour la première fois dans les toutes prochaines semaines, courant février, la Commission interministérielle d'octroi de la garantie de l'État pour examiner les premiers dossiers de demandes de garanties, il est très clair que nous avons besoin de dispositifs opérationnels pour s'assurer que soit des extensions soit de nouvelles constructions puisse voir le jour, faute de quoi, hé bien nous, ce serait un frein naturellement au développement du réseau, alors certes, la crise nous a obligés à à gérer l'urgence, mais je veux dire que tout au long de cette crise, nous n'avons pas perdu de vue l'objectif qui avait été assigné par le président de la République en 2018 et un certain nombre d'actions ont pu être conduite nonobstant cette crise sanitaire dans ce sens-là, je pense par exemple à la simplification de la procédure d'homologation, qui étaient engagés par le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports en lien avec, naturellement, les affaires étrangères et peut dire qu'il il a porté ses fruits puisque on dénombre 55 établissements de plus par rapport à 2018, donc on est au rythme d'une croissance d'une vingtaine de nouveaux établissements par an, je veux dire d'ailleurs que nous avons demandé à nos chefs de poste nos ambassadeurs, chacun dans leur pays avec naturellement l'ensemble des acteurs, de faire des feuilles de route véritablement pour structurer ce développement et s'assurer d'ailleurs que. Les extensions ou les nouveaux établissements ne viennent pas faire une concurrence directe à ceux existants, il s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, il s'agit d'y aller de façon ordonnée de façon cohérente et c'est donc le rôle qui est assigné également au réseau diplomatique de de ce point de vue-là et puis en matière de formation, nous ne sommes pas rester les 2 pieds dans le même sabot, nous avons créé le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger, le cap feu qui est proposée aujourd'hui aux étudiants se dessiner une carrière d'enseignant dans tous les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, les ISP et puis de nouveaux outils de pilotage ont été mis en place, il est vrai que certes au niveau des services à faire étrangères éducation se parlent régulièrement, mais je tenais absolument à ce que, au niveau des ministres aussi, il y a ce dialogue parce qu'on sait que parfois il y a des demandes de part et d'autre qui n'arrive pas à aboutir, parce que chacun campe sur des positions traditionnelles et à un moment il faut des décisions politiques pour avancer et donc le conseil d'orientation interministériel justement de l'enseignement français à l'étranger a été réunie sous l'autorité des ministres déjà il y a plusieurs mois, et nous allons poursuivre avec également ce nouvel outil. Voilà en quelques mots, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, l'ambition de cette proposition de loi et ambition que nous soutenons, qui s'inscrit pleinement dans les orientations qui sont les nôtres et dans les orientations que le conseil d'administration de l'AFE ajustement adopté hier puisque le conseil d'administration a adopté le contrat d'objectifs et de moyens 2021 2023 de l'agence, il y a eu donc une feuille de route stratégique et avec la proposition de loi qui vous est soumise, hé bien je crois que nous donnons à l'agence à l'ensemble du réseau, les moyens de se développer, de faire en sorte que cet instrument unique contribuent toujours plus au rayonnement de notre langue, de notre culture et de notre modèle éducatif dans le monde, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, dans la suite de la discussion générale, la parole est au président Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE pour 4 minutes, vous avez la parole monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le ministre, mais c'est le président de la commission des Affaires étrangères, il y a des gens des forces armées, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi est d'abord l'occasion de souligner l'excellent travail que fournit depuis 1990 l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, à travers les plus de 500 établissements homologués qui participent au rayonnement de la France et de la culture française,

se combiner le système éducatif à la culture locale a intégré et adapter l'école française au sein de nouveaux pays, les témoignages de ceux qui en c'est l'expérience le souligne cette et qui ont permis, d'un côté, la continuité du parcours scolaire d'un pays à l'autre pour les enfants de familles ce par exemple beaucoup

et que l'objectif n'est pas de les stabiliser à ce niveau, mais encore dans les armées, augmenter dans les années à venir, c'est pourquoi je comprends l'importance qu'il y a assuré une nuit représentation des familles et des anciennes élèves au sein du conseil d'administration, ceux qui sont passés par l'établissement de l'enseignement français à l'étranger, M. souligner leur attachement à leur souhait de valoriser sa raison d'école, même après l'avoir quitté, nous nous rendons aucune difficulté à se tenir l'ajout au sein du conseil à l'administration d'un représentant de associations d'anciens élèves de la cellule en France à l'étranger d'un représentant des associations de Français. L'nuit maternelle et bien renvoyé en temps de l'association nationale des écoles françaises à l'étranger, de la même façon, nous n'aurons aucune difficulté à voter en faveur de la création de 3 nouvelles missions, à savoir de contribuer à la formation des personnels. Le conseiller les promoteurs d'initiative de la conduite de leur projet d'homologation de l'établissement et d'instruire les dossiers de demandes de garantie de l'État pour financer les locaux d'enseignement, tout cela va dans le bon sens comme tout comme le fait de confier à l'agence, la gestion des instituts régionaux de formation et en tout cas, ici, on a bien fait de souligner que cet institut employeurs notamment pour objet de former les personnels et futur personnel il établissement de l'enseignement français à l'étranger, vous l'aurez donc compris le groupe RDSE votera pour cette proposition de loi peuvent apporter des améliorations dans la gestion de l'agence et dans le développement de l'enseignement français à l'étranger, il y vrai seront pas les carences bien il y a. Il est liée pour l'essentiel à des questions du budget du budget en encore, nous n'aurions pas pu examiner les dépenses du budget en décembre dernier, ce moment on met était mieux adapté qu'aujourd'hui, si pour mettre en valeur le travail des rapporteurs pour avis qui le projet de loi de finances, nos collègues, on a le grec et André Vallini je rappellerai certaines de leurs conclusions malgré la stabilité de la subvention allouée à la sa trésorerie reste il sera très sollicité, notamment pour venir en aide aux établissements en difficulté, ainsi qu'en faveur des États usant français au Liban, en même temps il faudra financer des opérations. Immobilière pour développer les capacités d'accueil des établissements malgré ces réserves, le groupe RDSE votera comme Janick et tout à l'heure cette PPL. Merci monsieur le président, la parole est maintenant Madame Hélène Conway Mouret pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la Commission et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais commencer par remercier notre collègue Samantha Cazebonne pour sa proposition de loi qui nous permet d'aborder les problématiques de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger l'AFE, au-delà des aspects purement budgétaire évoqué une fois par an lors de l'examen du projet de loi de finances, en effet, il s'agit d'un formidable opérateur public à la tête d'un réseau de containers qui, je le maintiens demeure unique au monde en ce qu'il n'est pas comparable dans son organisation, ni dans ses missions avec l'offre éducative, d'autres pays et qui continue à démontrer sa résilience dans la crise que nous traversons, il est l'un des principaux fleurons de notre diplomatie d'influence parce que, au-delà de notre langue, ce sont bien nos valeurs républicaines qu'il transmet cette proposition de loi poursuit 2 objectifs : le 1er de modifier la composition du conseil d'administration de la Uffe en y faisant entrer de nouveaux représentants d'associations en tant qu'expert et en doublant la représentation des familles cette évolution nous semble légitime dans la mesure où l'implication des parents d'élèves dans la gestion des établissements, tout comme leur participation financière sont croissantes, cependant, nous souhaitons que cet élargissement promeuvent la pluralité des fédérations d'associations de parents d'élèves, nous estimons également que la modification de la propension des sièges au sein du conseil d'administration ne doit pas se faire au détriment de la représentativité des personnels en effet le changement radical de modèle vers lequel veut tendre le gouvernement avec l'extension à marche forcée du réseau, par le biais d'établissements partenaires nécessiterait au contraire que leur soit donné un rôle plus important, nous souhaitons donc qu'à la fin de ce débat, l'équilibre prévu actuellement par le code de l'éducation soit rétablie, le second objectif vise la création des instituts régionaux de formation les IRF ayant vocation à prendre le relais des 16 établissements de mutualiser acteur de zones, il semblerait que l'AFE n'est pas attendu cette proposition de loi puisque le 1er IRF a été inauguré à Dakar, les 3 et 4 janvier dernier avant même son adoption cette précipitation marque sans doute l'empressement de la EFE à répondre à l'objectif fixé par le président de la République de doubler le nombre d'élèves, d'ici à 2030, il nous reste donc 8 ans qui implique, entre autres, d'augmenter le nombre d'enseignants formés, faut-il voir un changement de politique avec l'accélération de l'augmentation du nombre de personnels de droit local en effet le quinquennat s'est ouvert par des suppressions de postes d'enseignants conséquemment à l'annulation de 33 millions d'euros de la subvention pour charges de service public de Life en 2017 le nombre d'expatriés est ainsi passé de 1073 à 821 ETPT entre 2017 et 2021, soit une baisse de 21 % et de 5147 à 5004 résidant sur la même période soit moi 7 dans ce contexte, nous comprenons la volonté de renforcer la formation des personnels, afin de maintenir l'excellence et l'attractivité d'un réseau qui repose en grande partie sur la qualité de ses ressources humaines, recherché par les familles mais aussi sur des méthodes pédagogiques novatrices, nous interrogeons cependant sur le nombre et le statut des enseignants-formateurs qui seront déployés pour faire face à la demande, celle-ci pourrait s'avérer exponentielle du fait de l'ouverture de l'information, comme le suggère le texte d'une part à des personnels extérieurs du réseau qualifié ou non, et d'autre part au personnel exerçant dans les systèmes éducatifs étranger dans le cadre de la mission de coopération éducative fortement renforcée par ce texte. La question des moyens et de l'origine de ce-ci pour réaliser ses missions, c'est une activité économique, de formation, venait à être déployés mérite d'être précisé pour espérer accueillir à terme 700000 élèves, il sera nécessaire de procéder à une extension significative du parc immobilier de la greffe depuis 2011 : l'interdiction d'emprunt, handicap, l'agence pour conduire ses propres projets immobiliers dans ces établissements en gestion directe et créer des tensions croissantes avec les familles, sur lesquels pèsent lourdement l'essentiel de la charge ce point financier n'est certes pas abordé par le texte, mais si nous n'avons pas de salle de classe pour héberger et élèves et professeurs, il ne sert à rien de monter en puissance dans la formation de ceux-ci, à moins bien sûr que l'objectif soit de nous reposer intégralement sur le développement d'établissements privés, cela expliquerait que la Uffe soit en même temps, privé de moyens supplémentaires, humains et financiers pour remplir sa mission, en conclusion, le nombre d'amendements déposés, plutôt convergents, bien qu'issu le groupe politique différent montre que nous avons une autre vision que l'organisation future de l'enseignement français à l'étranger que celle proposée par le gouvernement, même si sur la forme, nous partageons les 2 objectifs de cette proposition de loi d'élargir la gouvernance et les prérogatives de l'agence si celle-ci répond aux objectifs du dernier contrat d'objectifs et de moyens et à un engagement pris auprès des associations de parents d'élèves, elle suscite de nombreuses questions et nous incite à ouvrir de futur débat sur un sujet qui nous tient tous à coeur, nous espérons que nos échanges cet après-midi, permettront de l'enrichir ce qui déterminera la position de notre groupe et je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant monsieur Joël Guerriau pour le groupe, les indépendants pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des Affaires étrangères et de la défense, mes chers collègues, je me réjouis que le prix Goncourt 2021 ait été attribué au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, cela met en valeur la langue française en démontrant qu'elle rayonne au-delà de nos frontières, la majorité de ses locuteurs vivent en effet en dehors du territoire national, alors 600 avec toute une variété d'accent et d'expression 220 millions de personnes parlent notre langue, et là, c'est bien sûr un atout dans le cas de nos échanges avec de nombreux pays, aux 4 coins du monde d'ailleurs, Monsieur le Ministre, vous auriez pu citer, parmi tous les auteurs que vous avez citées en préambule bien des échanges de biens d'autres mais des étrangers, cette fois-ci qui faire figure parmi les grands auteurs de notre littérature, y compris même parmi des Immortels de l'Académie française, notre réseau d'enseignement à l'étranger est un Avantage que nous devons préserver renforcer, il permet à nos concitoyens expatriés de bénéficier d'un enseignement dans leur langue maternelle, immergés dans leur culture cet enseignement contribue à partager le français et la culture française avec des étrangers qui le souhaitent aussi, nous devons assurer une évaluation permanente de l'efficacité de nos dispositifs, il y a 32 ans, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a été créé et 160000 élèves ont bénéficié en 2021 il y a 53 543 établissements et sur 138 pays, ce qui représente 375000 élèves, c'est important, le président de la République entend faire doubler les effectifs, et cette évolution nécessite bien sûr des adaptation et je salue le travail de notre collègue, Samantha Cazebonne qui nous propose d'en adopter certaines afin d'assurer une meilleure représentation, les fédérations de parents d'élèves, la proposition de loi leur offre de sièges supplémentaires, c'est une proposition qui a bien sûr beaucoup de bon sens, elle est complétée par la commission des Affaires étrangères par l'attribution d'un siège à l'association nationale des écoles françaises à l'étranger, sans voix délibérative, cependant il aurait été fort dommage en effet de se priver de la compétence et d'expérience de cet organisme présidé par notre excellent collègue Olivier Cadic l'agence aura une gouvernance plus équilibrée, ça a été dit, ce qui devrait lui permettent de mieux assurer ses missions actuelles, tout en se chargeant de nouvelles tâches. Il est impératif de renforcer la fait la l'enseignement français à l'étranger afin d'accroître et parfois de renouer l'influence française dans le monde, d'où l'importance de cette délibération pour soutenir les filières d'enseignement, les défis sont immenses, en effet, force est de constater que la francophonie est aujourd'hui menacée en Afrique des campagnes de propagande, 2 informations contre la France sont orchestrées par des puissances étrangères en Amérique du Nord, le wokisme pousse des instituts d'enseignement français à organiser des campagnes d'épuration littéraire comme ce qui s'est produit à Ontario, je le rappelle au Canada avec la destruction de près de 5000 livres en français à destination de la jeunesse, d'où notre fameux Tintin et Astérix, sans oublier le Moyen-Orient région stratégique pour la France, où plusieurs instituts d'enseignement français sont menacés de fermer à cause de conflits armés, une situation instable en Iran, en Syrie, et aussi malheureusement au Liban, la commission des Affaires étrangères, éclairé par le travail de notre excellent rapporteur a eu l'occasion de rappeler sa vigilance quant aux moyens financiers alloués à l'enseignement français à l'étranger alors que l'objectif fixé pour 2030, est très clair : l'évolution des financement l'est beaucoup moins un doublement des effectifs devrait nécessairement évidemment s'accompagner d'une augmentation significative du budget de personnel, nous nous réjouissons des ambitions qui sont nourris par la France pour que notre réseau à l'enseignement à l'étranger, continuer à rayonner et toujours plus, nous devons veiller à fortifier les piliers de notre action à l'étranger, la proposition de loi que nous examinons prépare sa montée en puissance, et bien sûr le groupe des indépendants votera avec enthousiasme cette proposition merci. Merci, cher collègue, merci. La parole est maintenant à monsieur Ronan Le Gleut pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit d'une part dans la logique du contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger la EFE pour la période 2021 2023 et d'autre part dans les orientations fixées par le président de la République d'un doublement du nombre d'élèves dans l'enseignement français à l'étranger d'ici 2030. En effet, la création de 16 instituts régionaux de formation ayant un statut d'établissements en gestion directe est une conséquence logique de l'augmentation des homologué d'homologation d'établissements ainsi davantage d'enseignants pourront être formés. De même la meilleure prise en compte de la voix des parents d'élèves, des parents gestionnaire au sein du conseil d'administration de la EFE des associations flamme français langue maternelle, la nef et des anciens élèves, les 600000 anciens élèves est une conséquence, elle aussi, à la fois logique et bienvenue pour ces raisons, il n'y a pas d'objection donc à adopter cette proposition de loi même si, lors de nos débats, certains amendements auront vocation à améliorer le texte, je pense notamment à le moyen qu'un conseiller des Français de l'étranger non membres de l'Assemblée des Français de l'étranger puisse siéger au conseil d'administration de la. Néanmoins, permettez-moi d'interroger la stratégie globale au regard des moyens alloués à cet objectif ambitieux et souhaitable de doublement du nombre d'élèves qui, au rythme actuel n'interviendrait pas avant les années 2005 En effet, un abîme existe entre les annonces et la réalité entre les paroles et les actes. Et cet abîme porte un nom : le en même temps. Source d'impuissance politique et de contradictions insurmontables. Vous dites que vous voulez doubler le nombre d'élèves et en même temps vous supprimez 512 postes d'enseignants, résidents ou expatriés et à peine arrivé au pouvoir en 2017 vous amputer le budget de la EFE de 33 millions d'euros et le rattrapage des années suivantes, n'a rien changé à une réalité que vivent les parents, à savoir que cette déstabilisation financière a entraîné malheureusement des hausses de frais décollage. Vous dites que vous voulez aider les parents à inscrire leurs enfants dans les écoles françaises à l'étranger et en même temps vous supprimez 10 millions d'euros pour les bourses scolaires, passant de 104 millions à 94 millions dans le programme 151 de la loi de finances pour 2022. Vous dites que vous voulez, accompagner les établissements scolaires et en même temps vous augmenter temporairement la PFC sa participation financière complémentaire, ce qui a entraîné des déconventionnement d'établissements scolaires. Vous dites que vous êtes auprès des écoles et en même temps vous créez une concurrence inéquitable entre établissements de nature différente, avec des homologations qui ne tiennent aucun compte de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire une carte scolaire. Vous dites que les établissements doivent se développer et en même temps vous empêchez les établissements en gestion directe les de recourir à l'emprunt et vous proposer une garantie de l'État pour les établissements conventionnés et les établissements partenaires qui est moins favorable qu'avec la nef, l'association nationale des écoles françaises de l'étranger. Je pourrais ainsi continuer, mais je crois que le message est suffisamment clair : votre politique est à la fois brouillonne et sans vision et cela nous désole étant un des 2 sénateurs désignés par notre Haute assemblée pour siéger au conseil d'administration de la mandat qui est évidemment bénévole, co-rapporteur pour avis du programme 185 sur la diplomatie culturelle et d'influence, mais aussi un Français de l'étranger, profondément attaché à notre magnifique réseau d'établissements scolaires partout dans le monde, réseau qui est un atout majeur de la France et que nous voyons, mise à mal ces dernières années, alors Monsieur le Ministre, je vous le dis solennellement mettait enfin en conformité vos paroles et vos actes sinon vous ne créerez que frustration et incompréhension et ce sera encore un échec. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Mélanie Vogel pour le groupe Écologie Solidarité territoire pour 4 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, chers collègues, la question de l'enseignement français à l'étranger, peu débattu, comme la plupart des sujets qui concernent les Françaises et les Français établis hors de France, cette proposition de loi nous donne donc l'occasion de prendre le temps, dans cet hémicycle pour aborder la question, est ce je crois en soi déjà un élément positif quel est le grand défi auquel l'enseignement français à l'étranger fait face, il y en a un, majeur, c'est une tension très forte entre des objectifs chiffrés extrêmement important, annoncé par le président de la République, doubler le nombre d'élèves à l'horizon 2030 et un abaissement des moyens fournis par l'État, c'est étrange quand on le dit comme ça, mais c'est ainsi, il y a une volonté politique de doubler le nombre d'élèves, mais elle n'est pas du tout corrélés à une politique visant à doubler les moyens mis en oeuvre par l'État en réalité en 2017, le gouvernement a même effectué une coupe de 33 millions d'euros entre 2016 et 2021 21 % de baisse d'effectifs pour les personnels expatriés et 7 % pour les résidents, le personnel de droit local croit 9 % les détachements aussi mais ça ne fait en tout cas un dixième du nécessaire. Comme la magie n'existe pas comme comment cet objectif de doublement du nombre d'élèves peut-il être rempli avec moins de moyens, est ce que c'est impossible, alors non, c'est possible, mais cela a un coût, un coût très fort en matière de solidarité et d'égalité de culture du service public et de traitements des enseignants, ça se fait mécaniquement, on s'oriente davantage vers un système guidé par des logiques privées ou le poids des frais de scolarité pèsent de plus en plus sur les parents, puisque la part d'engagement de l'État diminue et donc pour être plus précis sur les parents qui en ont les moyens, et où le statut des enseignants et de plus en plus précarisés pour faire des économies, c'est mécanique, à notre avis, au contraire, la logique de l'enseignement français à l'étranger doit être celle d'un service public afin d'assurer un enseignement inclusif de bonne qualité accessible et qui assure le principe républicain d'égalité des chances en conséquence pour les écologistes, plusieurs grandes réformes auraient pu être tout d'abord sur le réseau en lui-même, pour nous, la clé, c'est de renforcer la participation financière de l'État afin de juguler l'envolée des frais de scolarité, ça veut dire par exemple favoriser le recrutement d'enseignement d'enseignants titulaires, travailler à l'harmonisation des rémunérations et des avantages sociaux entre salariés de de droit français et contrats locaux, mettre en place des conventions collectives international et une charte sociale, de respect des droits des travailleurs et des travailleuses pour obtenir le Label EFE ensuite sur les bourses, les bourses a été dit, ont été amputées de 10 milliards d'euros pour nous, au contraire, ce qu'il faut c'est une augmentation substantielle du budget des bourses pour ne pas exclure une part de plus en plus grande de famille il faut par exemple modifier les barèmes d'attribution fixés en fonction de la situation économique et sociale de chaque pays pour réduire les inégalités, il faut une réforme du barème et des modes d'attribution des bourses pour les foyers monoparentaux et les couples séparés, dans ce contexte qu'est ce que fait cette PPL, bon, ça a été dit principalement 2 choses : assurer une plus grande représentation des familles et des anciens élèves au sein du conseil d'administration de la greffe et confié l'feu le soin de gérer les instituts régionaux de formation qui ont déjà été créés le 1er ayant d'ailleurs déjà été inaugurée en janvier, nous aurons l'occasion durant le débat sur les articles de discuter du contenu précis de ces propositions, mais vous l'aurez compris pour nous les écologistes, la priorité dans ce dossier, ça aurait été de réorienter structurellement notre modèle vers une logique de service public, c'est-à-dire une logique où prime l'égalité des chances, la qualité de l'enseignement, la mixité sociale de ces centaines de milliers d'élèves que nous avons vocation à accueillir, nous attendons donc avec enthousiasme les débats et les votes sur les différents amendements afin de déterminer si nous pourrons soutenir ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant madame Michelle Gréaume pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Monsieur Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission Défense, Affaires étrangères, monsieur le rapporteur. C'est-à-dire collègues cette proposition de loi nous permet comme trop rarement de débattre du réseau de l'enseignement du français à l'étranger, dans le fond, elle tente de répondre à deux enjeux majeurs le 1er est celui de la gouvernance, le réseau connaît une externalisation croissante ainsi sur le quinquennat si on dénombre 53 établissements de plus se Angers sur Direct diminue l'autre sujet d'inquiétude liée par ailleurs à l'importante l'importance prise par les établissements partenaires et l'augmentation des frais à poser aux familles ah si on parle en cumulé d'environ 5 milliards d'euros de frais de scolarité contre une subvention de 417 millions d'euros au réseau, avec des taux de prise en charge par les familles supérieures dans les établissements en gestion directe, comment, dans cette optique, et malgré les aides à la scolarisation espérer démocratiser l'accès à l'enseignement français à l'étranger d'ailleurs, si on peut se réjouir que les établissements accueillent une plus grande part d'élèves étrangers, certains parents craignent que l'AFE deviennent de plus en plus une machine à exclure les élèves français, qui représente aujourd'hui 37 % des effectifs au vu de ce contexte, la proposition de doubler la présence des représentants des familles au sein du conseil d'administration de la U. F. E est une bonne chose, avec la réserve toutefois qu'elle risque de restreindre la représentation des personnels, alors même que leur situation mériterait d'être examinée de près et améliorer, à ce titre-2 éléments me me viennent en tête tout d'abord l'augmentation massive et continue du nombre de personnels recrutés en contrats locaux bien moins protecteur, je m'interroge ensuite sur le choix fait par le réseau de refuser le versement de la prime informatique à ses personnels de droit locaux alors qu'ils ont été tout aussi sollicités que leurs collègues durant la pandémie. Dernière interrogation pour en terminer avec la gouvernance sur la perte Poutine intégrer au sein du conseil d'administration, un collège d'ancien élève à ce seul motif à ce seul motif, on a vu apparaître depuis plusieurs années maintenant des réseaux des anciens des alumni et autres associations, si ces dispositions mis en place par des anciens élèves ou les établissements eux-mêmes ont un intérêt certain sont-ils pour autant légitime à participer à la gouvernance des établissements. Peut-on imaginer que dans chaque conseil d'administration des collèges, lycées et universités siégeraient des élus supplémentaires dont la seule qualité d'avoir fréquenté l'établissement venons-en à la question des instituts régionaux de formation depuis le 1er janvier 16 d'entre eux ont été créés dans l'optique de renforcer la formation des personnels des établissements, c'est une mesure utile dans le contexte de l'augmentation espérée du nombre d'élèves, tout comme la proposition qui nous est faite d'en confier la gestion à la UFE, cela étant, je souhaite me faire une nouvelle fois les coûts des interrogations des familles,

quelles conséquences éventuelles sur les frais d'écolage déjà très élevé, y aura-t-il des conséquences sur le recrutement des personnels notamment Faut-il s'attendre à une mutation des fonctionnaires expatriés pour de nouvelles vagues de recrutement de droit local, y y aura-t-il aussi des conséquences sur le déploiement des personnels en place ou toujours nous espérer un remplacement systématique des enseignants, parti formé ou se former enfin quelle sera la place des investisseurs privés dans le processus, il faut-il voir une espèce de privatisation des gens engagés par ailleurs du réseau, toutes ces questions, sans remettre en cause le bien-fondé de l'idée même des instituts régionaux des formations interroge et tout en gardant en tête toutes ses réserves, notre groupe soutiendra la proposition de loi. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Olivier Cadic pour le groupe Union centriste pour 5 minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi déposée par notre collègue Samantha Cazebonne, dont je salue le travail et l'engagement en faveur de l'enseignement français à l'étranger. Vise à faire évoluer la gouvernance de la EFE il y a créé les instituts régionaux de formation, cette proposition de loi est destiné à soutenir le nouvel élan pour le réseau des écoles françaises à l'étranger, souhaitée par le gouvernement, qui cherche, entre autres, à développer le réseau actuel et accompagner la création de nouvelles écoles tout en associant mieux les familles à la vie des établissements. Comme le souligne notre rapporteur, les familles investissent largement dans les écoles. Il est juste, donc qu'elle puisse investir davantage dans l'administration du réseau, la proposition de loi, a justement pour objectif d'assurer un nouvel équilibre au sein du conseil d'administration de la EFE en attribuant 4 sièges au lieu de 2 représentants des parents d'élèves, tandis que les représentants du personnel en conserve 5 l'article 1er prévoit qu'un représentant des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger et un représentant des associations flamme français langue maternelle participe au conseil administration de la greffe en qualité d'expert. C'est une innovation qui semble faire consensus, je persiste à penser toutefois que les associations flammes qui propose à des enfants, des activités autour de la pratique du français en tant que langue maternelle ont une mission qui relève plus de l'institut français des alliances françaises que de la Successeur de notre ancien collègue André Ferrand, en qualité de président de la nef, l'association nationale des écoles françaises à l'étranger. Qui a tant fait pour l'enseignement français à l'étranger et je vous remercie, Monsieur le Ministre de l'avoir rappelé, je me réjouis de l'amendement, voté en commission qui permet de maintenir une représentation au sein du conseil d'illustration de la AFE dans la catégorie des participants en qualité d'expert. à la fin du mandat du président Hollande la Cour des comptes dénonçait un réseau d'enseignement fragilisé et invitait les autorités publiques à insuffler une nouvelle dynamique. Malgré le demi-milliard d'euros d'argent public consacrée chaque année. Le réseau de la EFE plafonné à 495 établissements scolaires fin 2017, soit moins que les 499 recensés à la création de la EFE 27 ans plus tôt. Pour mémoire, l'enseignement anglo-saxon compte désormais 9000 écoles qui scolarisent 5 millions d'élèves, elles sont donc près de 20 fois plus nombreuses que les nôtres aussi en décembre 2017 je me tenais à cette tribune exposait, devant vous mes chers collègues, l'urgence n'ont pas ambitieuse mais vital de doubler le nombre d'établissements dans lesquels l'enseignement français étaient dispensés. Pour éviter le déclassement de la France dans ce domaine, le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré le 27 mars 2018 à l'Institut français, nous allons développer les établissements partenaires avec l'objectif de doubler le nombre d'élèves accueillis au sein du réseau scolaire français d'ici à 2025 des pôles régionaux de formation seront créés pour former les nouveaux enseignants, fermez les guillemets. Même si l'objectif a été ensuite repoussée à 2030, j'ai toujours appuyé la démarche du président de la République qui a créé le nouvel élan que j'appelais de mes voeux. Nous pouvons nous réjouir que malgré la pandémie, le réseau est enfin entamer sa croissance en nombre d'établissements puisque, 3 ans après le discours de l'institut français à la rentrée 2021, ce réseau est désormais passé de 495 à 543 établissements scolaires homologué. N'en déplaise aux esprits chagrins, c'est un 1er succès qui marquera l'histoire du réseau et j'en suis sincèrement reconnaissant à Emmanuel Macron et à tous ceux qui ont contribué à ce résultat, la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui va permettent d'amplifier l'accroissement du réseau dans les années à venir pour atteinte l'objectif visé pour y parvenir, il faut recruter des enseignants en nombre, or nous savons que l'éducation nationale est incapable de nous les fournir à hauteur de nos besoins, cette expansion s'appuiera donc sur les enseignants recrutés en droit local, nous le savons, il faut donc former ces enseignants afin de maintenir le niveau d'excellence des établissements d'enseignement français, c'était le sens de la déclaration du président de la République à l'Institut français au sujet de la création des pôles régionaux de formation, elle se concrétise à l'article 4 qui prévoit que l'AFE gère également des IRF ces instituts régionaux de formation située à l'étranger et placé en gestion directe, qui assure notamment la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels exerçant dans le système éducatif étrangers cette formation indispensable des enseignants est une solution pour assurer l'attractivité des établissements. Qui permettra d'en augmenter le nombre et d'assurer le véritable rayonnement de notre réseau, ce qui freine le développement du réseau de l'enseignement français à l'étranger sont les meilleurs pourvoyeurs de clients des systèmes éducatifs étrangers lorsque j'ai été élu à Londres en 2006 le manque de place du lycée Charles-de-Gaulle nous amener à refuser 700 élèves chaque année, qui étaient redirigés vers l'enseignement britannique c'est pas ce que nous avons une politique d'expansion ambitieuse en créant 4 nouvelles écoles secondaires à Londres que nous avons pu mette fin à cette situation, le texte qui nous est aujourd'hui soumis nous propose de soutenir un nouvel élan et c'est bien un élan qu'il faut trouver cet élan dont nous avons un besoin impérieux pour reprendre une place et non la conserver dans le marché mondial de l'éducation international c'est bien en sortant du conservatisme qu'on pourra répondre à l'ambition du doublement du nombre d'élèves, d'ici 2030 et rêver d'un rayonnement, un peu plus éblouissant dans cette perspective stimulante revigorant d'un enseignement français à l'étranger, libre de croire de croître, pardon, le groupe centriste votera bien évidemment la proposition de loi, je vous remercie. Et chers collègues, enfin, dernier orateur Madame Else Joseph pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Si le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission de la défense, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à consolider tout un travail accompli depuis plusieurs décennies, pour renforcer notre présence éducative à l'étranger en 30 ans le nombre d'élèves a plus que doublé nos établissements sont reconnus et appréciés, il y avait donc tout un travail d'adaptation et de modernisation a mener à cet égard, l'amélioration de la gouvernance de la EFE est indispensable en raison de son rôle clé dans la présence de la France, en effet, au-delà de l'enseignement, c'est notre place dans le monde qui est en jeu, l'enseignement français contribue à notre rayonnement, il faut donc préserver cet atout. Je salue bien sûr les réformes envisagées pour la greffe et le travail de mon collègue Bruno Sido en 1er la meilleure prise en compte des parents d'élèves au conseil d'administration de la est indispensable, ils sont les premiers concernés et sont fortement impliquées dans le financement de l'enseignement à l'étranger. Il doit donc être mieux entendus et ce dont ont plus que leur expérience et leurs soutiens sont indispensables le rôle des familles doit être reconnu comme il en va, au sein de toutes communautés éducatives digne de ce nom, il contribue à l'image de nos établissements, de même les missions de la AEF feux ont été élargies, qu'il s'agisse de l'accompagnement dans les projets des nouvelles homologation de l'instruction des dossiers de demande de garantie de l'État, mais surtout de la formation des personnels qui exerceront dans les établissements d'enseignement français il faut former des enseignants mais aussi tout le personnel, à ce titre, je me réjouis de la mise en place d'instituts régionaux de formation, cela permettra de renforcer la qualité de notre enseignement à l'étranger, cette formation suppose évidemment une remise à plat en France, notre système de formation des enseignants, il n'y a que des cloisons étanches entre ce que nous faisons en France et ce que nous faisons à l'étranger, la griffe doit donc être un pilier dans notre rayonnement éducatifs dans le monde, mais il faut aller plus loin dans les moyens certes beaucoup a été dit, il y a un récent rapport d'information a même traité de la question, je salue mes collègues qui ont attiré l'attention sur ces différents problèmes car les moyens soulève de très grand, de très gros enjeu, comme je l'ai dit, c'est la question de la place de la France dans le monde qui est soulevée, notamment dans certaines parties du globe où se dessinent de nouveaux équilibres. Notre présence éducative est indispensable à notre présence économique industrielle et diplomatique, nous devons adopter une approche globale, car il est tout simplement question de la souveraineté de la France et de son rayonnement, nous devons éviter toute politique à courte vue, car c'est bien le long terme qui est en jeu ici, les 30 prochaines années seront tout aussi décisif que les 30 dernières. Notre enseignement est évidemment un marqueur de la francophonie, un marqueur fort de notre langue, un marqueur de notre culture, nos établissements sont des ambassadeurs estimé dans la défense et le rayonnement du français, c'est dire l'importance de l'enjeu, si nous voulons préserver la place du Français face à d'autres langues concurrentes, nous savons que la concurrence est féroce, agressive et ce qui se fait à l'étranger peut inévitablement rejaillir en France, il faut ensuite consolider la présence de notre pays par l'enseignement notamment dans des lieux stratégiques : comment faire pour que tout soit mis en oeuvre, au-delà des seuls effets d'annonce, à cet égard pour maintenir cette dynamique de consolidation l'AFE pourrait appuyer des projets de création d'établissements comme c'est le cas pour un lycée international à Taipeh, les porteurs de projets et les conseillers consulaires ont détaillé leur demande, ils sont prêts pour offrir à ceux qui le souhaitent une éducation en français à leurs enfants, former les enfants des Français installés dans la région à la langue française et pas seulement à l'anglais et aux Chinois comme l'environnement, il conduit notre langue est un précieux sésame, c'est pour cela qu'il faut permettre aux autres étrangers sur place, d'accéder à cet enseignement, c'est aussi ça le rayonnement de la France, on pourrait multiplier les exemples dont les demandes abondent de même comment consolider notre présence au Proche-Orient, la culture française, il bénéficie encore d'une aura, elle, peut-être une médiatrice dans les conflits de cette région un supplément d'âme parmi des cultures antagonistes à Simon dans le rapprochement des nations. D'autres projets pourraient donc voir le jour à la lumière d'une gouvernance de l'AFE améliorée. Le rayonnement du français dépasse en effet les seuls besoins de nos expatriés ainsi il faut aborder la problématique des parents qui ne sont pas français mais qui veulent donner à leurs enfants un enseignement en français et en français. Il faudra donc repenser le rôle de notre présence éducative à l'étranger, c'est urgent, bref, nous devons réfléchir sur les 30 prochaines années, parce qu'il faut aborder l'enjeu avec l'idée que notre place du XXIe siècle se joue aujourd'hui je tristesse avec les amendements approuvés par le rapporteur. Merci, cher collègue. La discussion générale est Close, nous allons passer à la discussion du texte de la commission. Avant l'article 1er je suis saisi d'un amendement 30 Monsieur Merci monsieur le président, le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se prive d'une extraordinaire expertise qui est l'expertise des conseillers des Français de l'étranger non membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, car en effet, Thierry 3 du code de l'éducation, alinéa 8 stipule bien que un membre de l'AFE et membre du conseil d'administration, ce qui est très bien, cela ne permet pas à l'AFE de désigner en plus un conseiller des Français de l'étranger non membres justement de l'Assemblée des Français de l'étranger et donc on se prive de ce réseau extraordinaire des élus locaux, des Français de l'étranger, on ne tient pas compte du changement de de la loi de 2013, notre collègue Hélène Conway Mouret qui justement change le niveau des élus locaux, les élus locaux, aujourd'hui les Français de l'étranger sont les conseillers des Français de l'étranger, contrairement à la situation antérieure, c'était justement les conseillers à l'AFP et donc cet amendement vise à à permettre à ce que ces élus locaux qui sont en contact, ce qui siègent dans les commissions locales des bourses scolaires qui sont en contact avec les parents d'élèves, les enseignants, les proviseurs avec toute la communauté éducative, hé bien qu'ils puissent avoir voix au chapitre au sein du conseil d'administration de l'AFE et que donc qu'un conseiller puissent siéger au sein de l'AFE c'est utile à la fois pour l'enseignement français à l'étranger et tout simplement pour la France puisque c'est le rayonnement de la France et sa volonté du doublement ça s'inscrit parfaitement dans la volonté de doublement du nombre d'élèves que cet amendement s'inscrit, je vous remercie. Merci, avis de la commission, monsieur le rapporteur. Voilà. Merci monsieur le président, la loi dispose que le conseil d'administration de la greffe comprend des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger, cette assemblée se compose de 90 conseillers élus parmi 442 des Français de l'étranger. Cet amendement introduit et le chiffre, un conseiller des Français de l'étranger, là où la loi fixe des grands équilibres ce qu'il y a introduit une incohérence sur cet amendement et plusieurs autres qui propose d'élargir le conseil d'administration de l'AFE, je suggère très modestement de nous en tenir à l'objectif de la PPL améliorer la représentation des parents d'élèves, à chaque fois que l'on ajoute un membre à ce conseil d'administration, il faut en effet aussi ajouter des autres membres notamment des représentants de l'État pour maintenir les équilibres en particulier la majorité de l'État, un conseil d'administration est une instance de pilotage non une assemblée représentative, s'agissant de cet amendement en particulier, il invoque la nécessité d'une représentation proche du terrain, il me semble que cet objectif est rempli, grâce à la participation accrue des parents d'élèves, les Français établis hors de France, ils sont également représentés par des parlementaires et par un membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, néanmoins la loi parle de représentants et non de membres de l'assemblée de française de l'étranger, dès lors, le décret d'application ne pourrait-il pas disposé et que cette assemblée peut désigner son représentant parmi l'ensemble des conseillers de Français de l'étranger, cela vous paraît-il envisageable, monsieur le Ministre, donc après la réponse de monsieur le ministre, je vous dirais que c'est une demande de retrait, sinon la vie serait défavorable. Oui, si je comprends bien, monsieur le rapporteur, vous dites après la réponse du ministre, mais quelle que soit la réponse du ministre ou demander le retrait bon alors Monsieur le Ministre votre avis.

être un conseil des Français de l'étranger, donc les conseils des Français de l'étranger sont bien représentés au sein du conseil d'administration de la greffe et et donc je crois que, finalement, l'amendement est satisfait du coup et donc cette effectivement je m'associe à la demande de retrait du rapporteur.

nos collègues souhaitent faire entrer au conseil d'administration et conseiller des Français de l'étranger supplémentaire auquel Madame Cazebonne ajoute une nuance puisque elle propose en effet que celui-ci sièges à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'Assemblée des Français de l'étranger alors comme l'a rappelé au Ronan Le Gleut ce sont des élus de de proximité qui siège par ailleurs à la commission locale des bourses sont généralement très impliqué dans les établissements scolaires de leur circonscription est également actif dans les associations de parents d'élèves et donc ils paraissent tout à fait qualifié pour apporter une expertise de terrain, je crois qu'il ne peut qu'enrichir les échanges lors des réunions du conseil d'administration et comme par ailleurs nous proposons un amendement qui permet de respecter les équilibres, nous pouvons en effet enfin en cas d'ajout de nouveaux membres au conseil d'administration, nous pouvons en effet ajouté un élu supplémentaire et pour cette raison, en groupe soutiendra cet amendement et celui de Madame Cazebonne à venir. Très bien, je mais aux voix l'amendement de 30 avec 2 avis défavorables qui est pour. Merci qui est contre. Moi j'ai 13 13, alors c'est un peu, bon, on va reprendre clairement qu'est pour lever bien la main. Qui est contre. Il est adopté,

proposée par l'article 1er ne correspond à aucune innovation puisqu'il est déjà possible d'inviter ces représentants au titre de leur expertise, il paraît adéquat pour, par exemple, les représentants des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger ou de l'association nationale des écoles françaises à l'étranger, en revanche, il nous paraît essentiel que les associations de français langue maternelle des flammes puissent participer de plein droit au conseil d'administration de la EFE étant donné le rôle primordial qu'elles sont amenées à jouer à l'avenir et je m'inscris en en faux à ce qu'a dit le sénateur Cadic lors de la discussion générale, de dire qu'elles ne font pas de cours de français que c'est du périscolaire, soit c'est une profonde méconnaissance de ce qu'elles font, ou au pire un profond mépris puisque il faut voir qu'il y a 170 associations dans 44 pays dont la mission principale, c'est justement d'enseigner le français aux enfants et adolescents vivant à l'étranger et scolarisés dans le système local, les écoles flamme faut savoir également qu'elles occupent une place croissante dans l'offre éducative française à l'étranger et à constitue un complément essentiel aux établissements homologués du réseau par ailleurs la constitution je récente d'une fédération des associations flamme à travers le monde dites fédération flamande leur offrent une nouvelle visibilité et une forte légitimité donc cet amendement, il vise à permettre à un représentant des associations de français langue maternelle de participer de plein droit au conseil d'administration de la EFE avec voix délibérative. Il y avait de la commission. d'une part, comme je l'ai indiqué précédemment, à chaque fois qu'on rajoute un membre du conseil administration à vrai dire on en rajoute 2 parce que l'État veut conserver sa majorité, par conséquent, on mettra un autre et, à vrai dire, si on écoute tout le monde parce qu'il y a d'autres amendements qui vont proposer la volonté première de l'augmentation de la représentation des parents d'élèves va diminuer et puis on en ajoute d'autres, donc les parents d'élèves vont réclamer à ce qu'on ajoute aussi. Bref, avec toutes les propositions qui sont là, on va arriver à un conseil d'administration qui pourrait, si les amendements adoptés comme le 1er qu'on a discuté à une quarantaine de membres au lieu de 30 ou 31 et donc c'est une perte d'efficacité, puis je voudrais quand même signaler mais ça a été dit par l'exposé de ce cet amendement. Que l'AFE que la flamme est représenté un expert technique avec moi, non de délibératives au conseil d'administration et par conséquent, peut-être qu'il ne votera pas, mais pourra dire ce qu'il a à dire,

Merci monsieur le président, moi je pense que compte tenu de la nature du réseau flamme qui est justement une multitude, une myriade d'associations et c'est ça qui fait sa force que justement, il faut respecter ce caractère associatif et il faut créer des synergies c'est c'est c'est l'idée donc de les associer comme expert au sein du conseil d'administration, mais je pense que justement la voix délibérative, quelque part, c'est de faire rentrer dans système ou potentiellement ils seraient régentées par d'autres que même, et donc je pense que vraiment, moi je suis très attaché au caractère associatif et donc l'association qui est prévu, à travers l'expertise au sein du conseil d'administration, enfin, en tant que membre expert est un est un un très bon mécanisme et je propose de donner sa chance au produit donc à ce stade, c'est un avis défavorable, défavorable, enfin, demande de retrait à défaut : avis défavorable sur votre amendement. Monsieur Leconte. Merci monsieur le président,

elle existe depuis 20 ans, ça a été une initiative de notre ancienne collègue Monique Cerisier-Ben Guiga, qui a lancé cette idée en 2001 et qui a permis à des Français qui vivent à l'étranger, de développer une socialisation en français de leurs enfants lorsqu'ils scolariser leurs enfants dans des écoles qui qui n'étaient pas des écoles françaises et c'est une démarche importante qui a pris de l'ampleur aujourd'hui et depuis déjà de nombreuses années, ceux-ci se fait sous la houlette de l'AMF. Mais elle ces missions sont d'abord l'enseignement français à l'étranger, or, à partir du moment où l'AMF a aussi cette mission de superviser les programmes flammes et en particulier les attributions des subventions flammes, il est important que le programme flamme ne soit pas la dernière roue du carrosse. Il est important que ce soit au coeur de la mission de l'agence et au coeur de son conseil d'administration et c'est la raison pour laquelle, pour les 20 ans du programme et je voudrais saluer la première association qui a fêté ses 20 ans un autre monde, hein, à Zagreb la semaine dernière et c'est les équipes qui le font vivre depuis depuis 20 ans, il est important que le conseil d'administration de l'avance. Aujourd'hui enfin mettent au coeur de ça, de, de, de ses préoccupations, ce programme flammes qui n'est pas la première mission de l'agence, mais qui aujourd'hui, après 20 ans, a besoin de ne pas être la dernière roue du carrosse et qui a besoin d'être au coeur des préoccupations et des arbitrages et des, des, des, des, des décisions de l'agence et c'est la raison pour laquelle cet amendement est important. Alors, allons-y, merci, je vous rappelle que le règlement est très clair : on parle de l'amendement on ne refait pas la discussion générale sur le caractère général de tous parce que sinon on s'en sortira pas cet après-midi, hein Madame Conway Mouret, vous vouliez dire ajouter quelques mots. Oui, c'est vraiment quelque mois Monsieur le Président, juste rajouter de de quoi je pense que, en effet, Monique Cerisier-Ben Guiga, qui est à l'initiative du lancement de de de flammes, il y a 20 ans serait très heureuse de voir l'évolution aujourd'hui de du du de ce réseau qui est absolument remarquable et de dire que nous avons tous été nous, élus locaux, je crois, l'initiative de la création d'un programme flammes dans nos circonscriptions respectives 2012, c'est au Sénat que les assises flamands ont eu lieu, ensuite j'avais demandé, dans une autre fonction à ce qu'un un espace ce soit dédiée sur le site de la UFE justement aux flammes et je crois que le budget qui est alloué cette année à ce programme montre que, hé bien ils méritent, en effet, toute sa place c'est pour ça que nous présentons et que nous soutenons cette cet amendement. Merci Madame Garriaud-Maylam. Oui, merci Monsieur le Président, 2 mots tout simplement pour rétablir une vérité, je suis désolé, le programme flamme n'a pas été créé par Madame Monique Ben Guiga, pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime, ça a été créé avant elle, il y avait déjà des petites écoles françaises aux 4 coins du monde, qui crée et avait été créée justement pour ce soutien aux français la langue maternelle, j'ai moi-même été à l'origine des tout premiers séminaires de formation des mamans pour pouvoir transmettre l'enseignement du français toutes les preuves sont là par contre effectivement madame Ghali Guiga a trouvé avec le groupe socialiste, le titre de flammes qui est effectivement une très belle appellation les ces écoles sont effectivement magnifique mais je voudrais revenir sur la question de la composition du conseil d'administration, cela fait 18 ans que je suis sénateur, j'ai même assisté à la création de l'EFE il y a très longtemps, il y a 32 ans lorsque j'ai été élu des Français, de Grande-Bretagne et d'Irlande à ceux qui s'appelait le Conseil supérieur des Français de l'étranger, mais je vous en prie, mes chers collègues, à chaque fois à chaque débat, chaque création d'institutions, on est toujours là, vouloir rajouter des postes dans les conseils d'administration pardonnez-moi de vous le dire, c'est souvent, on pense à ses électeurs, nous sommes élus au 2ème degré et je trouve ça extrêmement dommage parce que ce n'est pas l'honneur du Sénat, donc je voudrais dire une fois de plus, que je soutiens le rapporteur dans sa sagesse, nous devons limiter le nombre de membres de ce conseil d'administration qui deviennent pléthoriques et inefficaces, j'aurais dû le dire plus tôt lors de la discussion du 1er amendement mais mieux vaut tard que jamais, pour exprimer sa pensée. Oui, et puis une fois que ces 10, ça peut valoir pour toute l'après-midi, hein, allez, alors j'ai un coeur monsieur Cadic et s'il vous plaît, ne ne me remettait pas l'historique, sur 15 ans par les mois de l'amendement. Merci monsieur le président, pour l'historique, je remercie notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam, de l'avoir rappelé monsieur Chantrel écoutez mon cher collègue, il y a une différence effectivement que je ne méconnais pas entre l'enseignement français et l'enseignement du français et donc flamme, c'est l'enseignement du français, et c'est très exactement la mission qui est celle de l'institut français et des alliances françaises, donc je persiste à penser le leur développement serait mieux assurée si c'était dans le cadre de l'institut français et je ai connaît d'autant moins que quand on a lancé le plan école au Royaume-Uni, on a fait passer le nombre d'associations flammes de 15 à 50. Et je connais d'autant moins que j'ai même fait une proposition innovante pour leur financement, de mettre en place un chèque éducation et j'espère bien qu'on retravaille et qu'on supportera cette idole dans le futur mais puisque j'étais au conseil d'administration de la greffe en 2012 et que j'ai vu arriver les flammes. Dans la EFE à cette époque-là, je me souviens aussi que le budget qu'il aurait été alloué était de 700000 euros et que sous le président Hollande, il n'y avait plus que 300000 euros et donc voilà le ministre propose un 1000000 d'euros, il y en a qui parlent des flammes et il y en a qui faut. Allez, on va rester tranquille avec les flammes et je vais passer au vote maintenant donc sur un peu aller essayer ça je crois que tout le monde s'est expliqué pour savoir si Flame il y a l'amendement de 3 avec 2 avis défavorables qui est pour

Monsieur le ministre, la présente proposition de loi étant la participation au conseil d'administration de la AFE un représentant des associations dans ces élèves en qualité d'expert avec une voix non délibérative cet amendement propose d'associer également un élève actuellement scolarisés dans le réseau aux discussions du conseil d'administration, les lycées français ont en effet une représentation des élèves au sein des comités d'établissement et autres instances le vécu et les idées des élèves actuels permettrait une plus grande justesse dans la lecture de l'état du réseau merci. Merci, avis de la commission. Assurément, c'est une belle idée, mais est-ce vraiment l'intérêt de l'élève s'il paraît indispensable d'associer et les élèves à la vie des établissements, je m'interroge sur leur participation à une instance lointaine gérant des questions complexes budgétaire et caetera assez éloigné des préoccupations des élèves, une participation en visioconférence serait à tout le moins souhaitables, afin d'éviter à cet élève de devoir s'absenter de son établissement pour se déplacer à Paris ce qu'il y a un coût d'ailleurs quels élèves seraient choisis parmi les 370000 élèves en quoi représenterait-il l'ensemble des élèves du réseau de la maternelle au lycée, d'Europe et de l'eau. Année enfin etc, je vous propose une sagesse très défavorable. Avis du Gouvernement. Oui, demande de retrait à vie à défaut défavorable, les élèves y sont représentés dans les instances de l'établissement sur le terrain et il y a pas de structures représentatives des élèves au niveau du réseau à à l'inverse des autres parties prenantes, voilà ce qui explique que cette position, encore une fois, tenons-nous en à la représentation dans les instances des établis.

Qui est contre. Il est rejeté, le 21 Madame Cazebonne et là pour je dirais un peu le parallélisme des formes, puisque nous avons au sein de ce conseil d'administration de de députés, comme cela a été rappelé tout à l'heure de sénateurs également et puis moi je vous propose parce que il me semble que c'est quand même beaucoup plus simple à mettre en oeuvre la présence d'un conseiller français de l'étranger, mais membre de l'Assemblée des Français de l'étranger parce que je ne sais pas de quelle manière les les collègues qui ont proposé tout à l'heure, cet amendement envisage la nomination de ce Conseil français de l'étranger, mais à part inventer une nouvelle usine à gaz de la part, je dirais peut-être de l'administration qui va devoir beaucoup réfléchir à la méthode, je vous rappelle que les conseillers français de l'étranger sont répartis dans le monde entier, comment font-ils campagne pour ce poste, je trouve que il était un peu hasardeux de se lancer dans dans un tels amendements alors que nous avons une instance qui représente ses conseillers français de l'étranger et dont l'organisation pour mettre et nommer un membre du conseil d'administration est déjà connu, je trouve que la facilité nous amène effectivement à défendre cet amendement et et faciliter aussi la vie de l'administration, par de la même.

2 Français de l'étranger au conseil d'administration et puis. Et, par conséquent, puisque monsieur le président, ma dit de ne pas répéter ce que j'ai déjà dit je suis défavorable. En réalité, ce n'est pas du domaine de la loi, c'est du domaine réglementaire et moi je souscris à l'idée que nos élus locaux soient soient mieux représentées, je l'ai dit, je pense que c'est mieux que ça passe passe à travers un conseil des Français de l'étranger qui siège à l'AFE et qui est effectivement cette homothétie entre les départ les les députés et les sénateurs et les conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger, donc c'est une une sagesse positive enfin une demande de retrait puisqu'en fait c'est du niveau réglementaire et donc je j'ai entendu l'appel de de de Samantha Cazebonne que je reprendrais volontiers par voie décréta l'est et au motif de cet engagement, je vous propose de retirer l'amendement. Madame Cazebonne, monsieur le ministre. Je sais que vous avez tenus tous vos engagements jusqu'à présent pour cet enseignement français à l'étranger, donc je je retire mais au bénéfice évidemment de votre engagement. Je mais on voit l'article 1er qui est pour. Qui est contre. Il est adopté la gouvernance de l'Agence pour l'enseignement des Français à l'étranger, le type de cette proposition de loi laisse présager des changements majeurs dans la composition du conseil d'administration de l'agence, et donc de nouvelles orientations, or dans les faits, il n'en est rien l'AFE est aujourd'hui administrée par un conseil d'administration, comprenant un président de députés, de sénateurs et des membres répartis en 2 collèges le 1er représentant au moins la moitié des sièges est composé de représentants du gouvernement, le second composé de moi pour moitié de représentants du personnel est également constitué de représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements et des fédérations d'associations de parents d'élèves, cet article 2 propose de modifier uniquement la proposition à l'intérieur du second collège afin d'augmenter la représentation des parents d'élèves et de minimiser celle des représentants du personnel, cette modification n'est que cosmétique puisqu'elle ne change en rien l'équilibre au global du conseil d'administration, où les représentants des ministres restent majoritaires, ces derniers continueront d'entériner des propositions qu'ils ont fait, sans que le second collège ne puissent finalement faire entendre sa voix, la répartition actuelle ainsi que celles que proposée par cet article, prive le conseil d'administration de toute collégialité et relègue les membres du second collège au rang de spectateur impuissant, afin que le Conseil devienne un véritable organe stratégique, il faut avoir le courage et la confiance de laisser les auteurs du réseau que ensemble les personnels et familles décident de l'avenir de l'agence cette ambition est celle que je porte dans l'amendement que je défendrai. Merci le 31 madame Vogel. Oui merci monsieur le président, donc, cet amendement propose la suppression de l'article 2 l'article de modifier la composition du conseil d'administration au bénéfice des parents et au détriment des personnels enseignants, ce changement, ça été explique qu'il y a un peu dans la déclaration générale mais ne nous paraît pas judicieux parce que nous sommes à un moment où nous manquons d'enseignants et où nous avons une logique politique qui consiste à faire peser de plus en plus le le coût le coût de la scolarité sur les parents et que, au fond, maintenir la représentation des personnels peut au contraire contribuer à éviter, du moins contenir cette dérive qui va vers une logique plutôt de marcher à l'inverse d'une logique que nous défendons davantage qui est une logique de service public, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, cet amendement, c'est rien moins que de supprimer l'article 2 ça va complètement contre, c'est absolument radicale, tout à fait, Monsieur le Ministre, et à vrai dire, les nouveaux équilibres introduit par la proposition de loi doit fermer de passer les représentants des parents d'élèves de 2 à 4, ce qui est normal, tout le monde est d'accord, et par conséquent jamais la commission a émis un lit défavorable Oui, même avis juste pour dire donner l'évolution de la contribution des parents un enseignement français à l'étranger en 2007, ils représentaient 70 % du financement de l'enseignement français à l'étranger et on en est aujourd'hui à 80 % c'est-à-dire que sur 2 milliards 5 tout l'État met 500 millions d'euros, les familles, mais 2 milliards d'euros, je pense que c'est bien de reconnaître cet engagement qui va d'ailleurs au-delà d'un engagement financier qui est aussi un engagement moral au quotidien et donc le fait qu'on tienne cet engagement qui a été pris de doubler leur représentation, donc avis défavorable sur l'amendement de suppression. jeu mais aux voix l'amendement 31 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté, le 23 Madame Renaud Garabédian, vous l'avez en partie présentée dans votre intervention. Merci monsieur le président je pas reprendre la composition du Conseil pour que le conseil d'administration de la FAO devienne une instance stratégique de débats et de réflexion, cet amendement propose que les représentants des ministres occupent moins de sièges au conseil d'administration de l'AFE merci. La commission. Alors un conseil d'administration n'a pas vocation à être seulement une instance de débat et de réflexion, c'est une instance de pilotage d'orientation et de décision, il n'existe pas de libre administration des établissements publics, si ceux-ci disposent d'une autonomie, il reste un prolongement de la personne publique à laquelle ils sont rattachés, qui exerce sur un pouvoir de tutelle, on ne peut pas éluder l'existence de ce pouvoir de tutelle qui est un pouvoir d'approbation ou d'annulation des décisions prises la majorité dont l'État dispose au Conseil des et le pendant logique de l'exercice de la tutelle et donc l'avis défavorable. Qui est contre, il est rejeté. Un amendement et un sous-amendement le 35, monsieur le rapporteur. ce sous-amendement soulève légitimement la question de la représentativité des fédérations d'associations de parents d'élèves qui tient monsieur le rapporteur. Je vous demande pas de donner votre avis sur le sous-amendement qui vient mais de présenter l'amendement de la commission le 35.

l'article 2 a pour objectif d'assurer non lieu représentation des élèves au conseil d'administration de l'cet objectif est légitime, comme l'a dit Monsieur le Ministre, les de la finance 80 % environ de l'enseignement français à l'étranger, la réforme proposée permettra donc d'assurer la présence de quatre présentant l'augmentation du nombre de représentants des parents pose la question de la mesure de la représentativité des fédérations d'associations de parents d'élèves, les 2 fédérations actuellement représentés sont la EFE et sont reconnus d'utilité publique et dispose d'une légitimité incontestable, il conviendra de s'assurer que les fédérations représentées continueront toute à disposer d'une légitimité suffisante d'éviter la présence de fédération marginal ou à vocation purement locale, tout en permettant aux parents d'élèves d'être aux parents d'élèves d'être représentés dans leur diversité, cette d'amendement met donc l'accent sur la notion de représentativité, sans se prononcer sur les critères de représentativité qui reviendra au au gouvernement de fixer par décret. Merci alors votre amendement et sous-amendé par Madame Cazebonne, au nom de la commission des affaires étrangères, Madame Cazebonne, le sous-amendement 39. Merci Monsieur le Président, alors moi je vais évidemment dans le sens du rapporteur qui finalement pose un sujet essentiel sur la Table puisque nous allons voter pour augmenter le nombre de sièges des des représentants des parents d'élèves, ce qui est important, vous savez, notre notre réseau et plurielle, il est très vaste. Avec des zones géographiques très diverses et avec donc des problématiques aussi très diverses, donc je je je souscris totalement au fait qu'il faut qu'elle soit, cette représentation des parents extrêmement représentatif pour le coup, mais, mais, moi, si vous me permettez, j'aimerais ajouter un point parce que je crois qu'il y serait assez inopportun pour ce réseau de voir pulluler un peu un certain nombre de de représentation qui s'auto-désigneraient à travers le monde donc je je crois qu'il y a un critère de stabilité intéressants que je vous soumets mes chers collègues, serait qu'a minima, ces fédérations puisse être reconnue d'utilité publique fin par le biais d'associations évidemment mais reconnue d'utilité publique, ce qui je pense, donnerait un gage d'assurance, là aussi, puisque durant 3 ans, ils doivent démontrer de la stabilité de leurs effectifs et d'un certain nombre de critères, donc je pense que ce point là pourrait être intéressant à entendre pour différencier les différentes associations et leur représentation au conseil d'administration. Voilà, merci, merci, alors, avis de la commission, cette fois-ci sur le sous-amendement 39 avant l'avis du gouvernement sur les 2. les critères de représentativité proposées sont très exigeants, même après la rectification opérée par Madame Cazebonne, tendant à ce que les fédérations soit simplement reconnue d'utilité publique, par conséquent, la proposition de loi conduirait donc probablement à la désignation de représentants supplémentaires de ces fédérations déjà représenté vaudrait-il pas mieux chercher une meilleure représentation de la diversité des parents, je vous propose d'en rester à mon amendement répondant d'une façon plus souple à la question ici posée de la représentativité de fédération d'associations de parents d'élèves et par conséquent j'émets un avis à titre personnel parce qu'on n'a pas vu cela en commission un avis défavorable. Alors, avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement favorable à l'un et à l'autre. Favorable aux 2 bon oui monsieur, allez-y, Monsieur le comte. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues évêques non c'est un sujet important, à partir du moment où on lui dit on, on augmente le nombre de représentants des associations de parents d'élèves, toutefois, monsieur le rapporteur, même si Jean nous pourrions souscrire à votre amendement sur la question de la représentativité, la question est de savoir comment est-ce que le gouvernement et le peut-être que Monsieur le ministre, si pourrait nous éclairer quand est-ce que le le gouvernement et estime utile et et comment mesurer la représentativité des, des, des, des, des différentes associations, sachant que, dans chaque établissement, les parents d'élèves sont représentés dans les conseils d'établissement compte tenu de la circulaire vie scolaire qui définit la manière dont les les parents sont élus le le le le ministre compte tenu de l'évolution du nombre de de parents d'élèves, vous comptez vous appuyez sur les élections aux conseils d'établissement et la filiation des parents aux différentes associations de parents d'élèves pour mesurer la représentativité, c'est un point important parce que si nous avons l'assurance. Que le gouvernement prendra en compte la représentativité des associations de parents d'élèves sur la base de la circulaire vie scolaire et des élections au conseils d'établissement alors effectivement l'amendement de de notre collègue rapporteur un sens. Alors, je vais mettre aux voix non monsieur le comte, vous n'avez pas interpeller le ministre donc je vais mettre aux voix. Alors c'est un peu ennuyeux parce que le rapporteur est bien d'accord, il a donné un avis défavorable au sous-amendement. Je mets donc aux voix d'abord le sous-amendement le 39 avec un avis favorable du Gouvernement défavorables du rapporteur qui est pour le sous-amendement. Qui est contre. Il est rejeté, je mets aux voix maintenant alors l'amendement non sous-amendé, on est bien d'accord. C'est l'amendement de la commission avec avis favorable du gouvernement qui est pour.

Oui, ben je vais défendre indirectement le le 4 je je vais retirer le 5 pour une raison très simple, c'est que le le IV est un amendement de cohérence qui prend justement en compte ce que notre assemblée a décidé, en accordant un siège supplémentaire au sein de l'agence à travers un élu un moment il il vise justement à rétablir la proportion des représentants des personnels enseignants, sans empêcher l'augmentation des sels de des parents d'élèves désormais inscrite dans le marbre, c'est pas compliqué, c'était un peu la le problème de ce texte initialement, c'est que la l'augmentation de la présence au sein du conseil d'administration, des représentants des parents d'élèves se faisait au détriment des personnels et plus particulièrement des enseignants, le sexe ce gouvernement de traite pas bien les enseignants mais ça devient une obsession sur tous les textes avec que vous pouvez vous tapez sur les enseignants, donc je pense qu'il est essentiel de pouvoir garantir ce thème cette présence telle qu'allait. de de d'un équilibre qui est possible, c'est-à-dire que les 2 étaient possibles, on pouvait très bien augmenter le nombre de personnels, des parents d'élèves, enfin, les parents d'élèves et le personnel enseignant et c'est ce que permet cet amendement merci. Merci à l'avis de la commission, on est bien d'accord, uniquement sur le 4 le 5 est retirer donc avis de la Commission sur le 4 E. Oui, monsieur le président je veux bien suivi cet amendement devrait logiquement être retirés car il suppose l'adoption du numéro 3 de l'article 1er qui n'a pas été rejetée par conséquent il reste effectivement l'amendement réduit à un quart la place de fédération d'associations de parents d'élèves plutôt qu'un tiers, et par conséquent c'est une demande de retrait sinon avis défavorable.

Alors que le président de la République annonçait au printemps 2018, sa volonté de voir le nombre d'élèves doublé dans le réseau à l'été, le ministère des Finances a bloqué le dispositif de la nef, qui permettait d'obtenir des garanties de l'État, un dispositif qui a permis de développer, d'aider, de faire 190 prêtre pour 112 écoles au cours de son existence, avec encore 50 près qui sont actuellement en cours jusqu'en 2047, le nouveau dispositif qui a été votée. En décembre 2020. Compte tenu des de de sa mise en oeuvre et compte tenu de de sa non-opérabilité. N'a pas encore permis d'aider un seul établissement scolaire. Et une raison est clair. C'est que le coût de cette nouvelle garantie de l'État peut-être prohibitif puisque c'est Bercy qui fixe le montant de la provision qui doit être versé pour rémunérer la garantie de l'État

par an à verser alors que, avec le dispositif de la nef, ceci était entre 03 et 04 % par an, ce qui donne la garantie, une garantie de l'État totalement ineffectives voilà, Monsieur le Ministre, résultat de votre politique, plus aucun établissement depuis l'été 2018 est en mesure de demander une garantie de l'État opérationnel et à un tarif acceptable alors. Nous proposons par cet amendement au minimum et par transparence, le fait que le conseil d'administration. Donne un avis sur le montant de la provision que l'État demandera lorsqu'il donne sa garantie à un projet immobilier. Avis de la commission. a mis en place le dispositif de garantie qui se substitue à l'association nationale des écoles françaises de l'étranger l'année. Ce nouveau dispositif est hélas moins favorable que le précédent, comme il a été dit, il prévoit en particulier une rémunération de la garantie par une commission variable en fonction des risques encourus, alors que cette commission était auparavant unique et mutualisé, elle était de 0 4 dans ce contexte de la proposition de loi donne à la UFE un rôle d'instruction des dossiers de demande de garantie de l'État, elle joue donc déjà un rôle d'expertise qui sera utile pour déterminer les taux de la commission, le taux de la commission, mais serait-elle bien dans son rôle vis-à-vis des établissement en donnant formellement un avis sur ce taux qui sera de toute façon déterminée par le ministre chargé de l'économie, je crains que cela ne la mettent dans une situation délicate aussi, la commission a émis un avis défavorable Même avis monsieur le président, en précisant en fait que la UFE sera bien impliqué dans l'instruction du dossier puisque son service immobilier sur le service du développement le SDR justement participera à la à la vie données sur le dossier après que le conseil consulaire dans le pays concerné également été que le chef du poste diplomatique est soumis le dossier à la EFE donc l'avait fait pleinement partie prenante dans l'élaboration du dossier hé bien, on passe à la Commission interministérielle et j'y serai particulièrement vigilant puisque, avec le double rattachement désormais Bercy et Quai d'Orsay, donc je pense que ça pourra peut-être contribuer naturellement la chose et sur le le taux, je veux dire que le taux peut-être aussi entre 0 32 et 1 8 mais il peut avoir des taux à 0 32 à 0 40, donc ce qui pouvait être équivalent à ce qui était fait auparavant par la nef et vous savez que si on a été amené à à à à faire évoluer la nef, c'est que, aussi, au regard de ses activités, il n'était pas banal que une association est une activité qui s'apparente à une activité bancaire, il est temps, je crois, localisé dans cette même institution.

et je dois dire que dans le cas de mes activités, j'ai, j'ai eu recours et fait une demande d'ailleurs à ce dispositif, dont je salue l'an l'engagement d'André Ferrand, qui a toute mon amitié sur sur le sujet et évidemment aussi à Olivier Cadic qui aujourd'hui a pris sa succession, voilà, je crois que le le ministre l'a rappelé le le. Cadres et c'était admis par tous, aussi, était à la limite, nous allons le dire ainsi de de la légalité, il fallait absolument, il y a apporté une réforme je crois que cela a été fait, la nef aujourd'hui a toute vocation à se renouveler, a proposé de de nouveaux services justement pour pallier à ce différentiel mais je vous rappelle quand même cher collègue que désormais c'est l'État directement qui garantit, je pense que ce point là n'est pas négligeable et et lorsque nous sommes dans une logique aussi comptable, je pense que ce sont des points qui ne peuvent pas échapper non plus à votre vigilance, de s'assurer effectivement même si la nef a toujours bien gérées, il faut le reconnaître et il faut même le saluer, hé bien malgré tout aujourd'hui, il y a des cadres réglementaires à respecter, et moi je souhaite en tout cas, bonne chance à la nouvelle à 9. En tout cas et je, je, je, j'espère qu'elle sera aussi apporter de de nouveaux services à cet enseignement français à l'étranger. Naturellement, Monsieur le comte je je le redis une dernière fois, après quoi j'appliquerai le règlement à la lettre l'amendement seulement l'amendement, vous n'avez pas à sortir de l'amendement pour faire une discussion générale

Entre 2018 et aujourd'hui il n'y a plus une seule garantie, l'État qui a été attribué. La nef a particulièrement bien gérées. Dans la mesure où. il n'y a pas les les défaillances qui ont pu exister, ce sont des défaillances qui ont été régulé par la mutualisation du risque au sein même de la MNEF. Donc le fait de changer les choses et de ne pas permettre aujourd'hui alors que le dispositif a été votée depuis plus d'un an que un nombre important d'établissements attendaient le nouveau dispositif que un an après, aucun établissement n'est plus demandés n'ait pu mettre en 9 ce dispositif montre bien que ce nouveau dispositif ne fonctionne pas que votre politique ne fonctionne pas et pourquoi, parce que le coût de 1 virgule 8 et totalement impossible. 1,8 % du montant engagé c'est juste : impossible pour les établissements qui ont justement besoin de la garantie de l'État. Mais oui, mais c'est parce que justement votre il y avait beaucoup plus de, de, d'établissements qui attendait le nouveau dispositif si un an après, vous n'avez toujours pas donné la garantie de l'État, c'est bien parce que le dispositif n'est pas opérationnel et est trop élevé aussi je vous incite aussi à monsieur le rapporteur, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette proposition les taux doivent être publics. De manière à ne pas bloquer. Et, de manière à permettre le développement des établissements. Si nous voulons le développement du réseau, il ne faut pas faire payer cher la garantie de l'État dans les pays où justement s'il n'y a pas de garantie, on ne construit rien parce que justement dans ces pays-là, les taux d'intérêts sont élevés.

Qui est contre. Il est rejeté, monsieur Leconte le 6. Merci monsieur le président, toujours dans cette volonté de d'assurer un un développement du réseau et comme notre rapporteur l'a signalé l'agence depuis de nombreuses années et là ce n'est pas une nouveauté du gouvernement actuel, c'est malheureusement depuis depuis longtemps. N'a plus la capacité d'emprunt toutefois lorsqu'on regarde le code de l'éducation sur la sur qui et qui porte qui donne, elle donne bien le code de l'éducation donne bien. La prérogative à l'agence de lever l'emprunt. Il est quand même étonnant qu'une fois que cette prérogative de lever l'emprunt et dans le code de l'éducation dans la loi. Parce qu'une autre loi. Donne une prérogative au gouvernement de décider qui est Hodac.

repose la question repose la question de la réalité. De ce que nous, on nous dit depuis des années. C'est-à-dire que est-il réel que l'avait fait, n'a pas de capacité d'emprunt alors que dans la loi, c'est indiqué qu'elle peut lever l'emprunt. Et nous souhaitons réaffirmer que la greffe peut lever l'emprunt et que elle peut lever l'emprunt après examen de son conseil d'administration. Que la loi soit respectée et que le gouvernement respecte la loi, qu'à partir du moment où, dans le code de l'éducation, nous avons déjà voté au Parlement que l'AMF pouvait lever l'emprunt, nous souhaitons que l'avait fait, puissent le faire et que ce soit sous contrôle de son conseil d'administration, c'est ce qui permettra le développement du réseau. Alors, lors de la création de l'AFP, il est effectivement prévu qu'elle puisse emprunter, mais la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 a interdit aux Hodac d'emprunter. Et j'ouvre les guillemets, je reprends le texte nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables ces Hodac sont au nombre de 700 avec la on imagine que si chacune emprunter pauvreté qui est déjà submergé par les dettes, il n'en sortirait plus il y a cet amendement n'apporte pas de solution à cette situation, il ne permet pas de remettre en vigueur la disposition implicitement abrogées par la loi de programmation des finances publiques, seule une loi de fil financière pourraient le faire et encore à l'initiative du gouvernement, le dispositif proposé et donc inopérants, l'avis est défavorable. Avis du Gouvernement.

et donc l'Insee en date de mai 21 je lis il est exactement ce qu'elle nous dit le comptable national considère ainsi que la UEFA est une administration publique appartenant du fait de sa compétence au sous-secteur des administrations centrales et classé sans ambiguïté dans le secteur des donc voilà les choses sont claires de ce point de vue là maintenant, c'est vrai, s'était excellemment dit la décision a été prise en 2011 de 2011 à 2014, vous aviez une majorité au Sénat, vous aviez une majorité absolue national Hélène Conway Mouret a été ministre, que ne l'avez-vous fait. Monsieur le comte brièvement parce que vous n'avez pas monopoliser la parole tout l'après-midi. Monsieur le président, nous examinons une loi, je suis désolé, il y a des amendements les on les discute, monsieur le Ministre, j'ai bien précisé. Que c'était pas la faute de votre gouvernement, donc c'est pas la peine après de de nous titiller, je le sais parfaitement. Bon, ceci étant dit, monsieur le rapporteur, vous êtes parlementaire. Monsieur le rapporteur, vous êtes parlementaire quand une loi. Précise que l'AMF a une capacité d'emprunt. Acceptez-vous derrière que le pouvoir réglementaire place l'AFE.

Et ce n'est pas une question d'attaques de telle ou telle gouvernement je dis c'est aujourd'hui, en tant que parlementaires, nous avons voté la loi, il n'est pas logique. De se faire dessaisir par une procédure opaque. De qui décide. De qui est placé en Hodac surtout Monsieur le Ministre. Que elle avait fait, aujourd'hui, on peut le regretter, mais il y a des recettes qui sont plus des recettes qui viennent de son activité qu'une subvention publique.

Donc 2 raisons : la première, il n'est pas logique qu'en tant que parlementaires, nous acceptons que le pouvoir réglementaire retire. Le pouvoir que nous avons quelque chose que nous avons voté dans la loi et la 2ème chose c'est que même si nous acceptons le principe des

j'juste si dans l'esprit, je, je, je pourrais rejoindre mon collègue parlementaire, je voulais simplement dire quand même, pour établir aussi une vérité que ce n'est pas satisfaisant, ce que je veux dire je, j'en conviens mais c'est quand même une réalité aujourd'hui l'agence d'enseignement français à l'étranger, à quand même recours à un emprunt qui est octroyée par France trésor qui a des dérogations pour aller jusqu'à sept parfois 9 ans, de capacité de remboursement donc je j'entends et et j'aurais tendance à vous rejoindre sur le principe on nous sommes d'accord malgré tout il y a quand même une possibilité d'emprunt par dérogation qui est accordée à l'agence. Très bien, je mais aux voix l'amendement 6 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Il y a rejeté monsieur Leconte on ne pourra pas dire que vous manquez de temps de parole l'amendement 7. Merci Monsieur le le président, cet amendement vise à offrir une lisibilité une stabilité aux établissements français à l'étranger quand alors là à aux participations qu'il qu'il reverse à l'agence en 2017, par exemple, cuite à une coupe de 33 millions d'euros de subventions publiques en quelques semaines, l'agence a de a augmenté de 50 % sa demande de participation financière complémentaire aux établissements conventionnés. Ce qui est juste ingérable pour des établissements qui veulent et qui ont besoin de prévisibilité. Nous savons aussi que l'agence aujourd'hui envisage, compte tenu de l'absence de gros financements publics à la hauteur de ses ambitions, une changement changement dans la participation des établissements, de manière à ce que, comme on dit en novlangue ce soit plus dynamique, c'est-à-dire en fait que ça augmente tous les ans, sans avoir besoin d'en changer les paramètres, il nous semble logique. Que les demandes de participation que l'agence formule auprès des établissements scolaires. Soit normé transparents et discutées par le Conseil d'être, d'administration, c'est la raison de cet amendement. La loi se borne à indiquer que l'agence est administrée par un conseil d'administration, les domaines dans lesquels le conseil d'administration de l'hiver sont fixées par décret en l'espèce l'article D. 452 tiré 8 du code de l'éducation, dispose que le conseil d'administration délibère sur les principes selon lesquels sont déterminées les redevances des rémunérations de toutes natures, perçue par l'agence et donc l'avis est défavorable.

Merci monsieur le président je vous rassure, c'est la fin de votre supplice parce qu'après c'est beaucoup d'un mois d'amendements à défendre d'abord je voudrais commencer cette prise de parole en rendant un hommage au aux enseignants du réseau et à l'ensemble des enseignants qui exercent en France et pour la France. Nous savons aujourd'hui que nous avons énormément de difficultés à. à les recruter, compte tenu du niveau de leurs rémunérations, en particulier et à l'étranger, il est dommage qu'un certain nombre de personnes qui exerce de manière en recrutement local ne puisse opérer ne puissent avoir le choix d'être titularisé en restant à l'étranger, je voudrais rappeler quelques éléments nous le président de la République en 2018 à à à signaler avant sa volonté de voir le nombre d'élèves doublé entre 2018 et 2030 dans le réseau, pourtant les moyens qui ont été attribués, si on le rappelle, c'est cruel entre 2017 et 2022, on est passé de 6169 à 5609 en terme de plafond d'emplois pour les titulaires, placé auprès de l'greffe la croissance des moyens 397 millions en 2017 à 420 en 2022, voilà comment voulez-vous. Faire plus. Avec moi, en maintenant la qualité, alors bien entendu, dans ce cadre, les instituts régionaux de formation auront leur utilité. Mais s'il faut le dire. Ce sont les parents qui financeront ces nouveaux instituts régionaux de formation parce qu'il n'y a pas de moyens nouveaux. Il n'y a pas de moyen nouveau. Il n'y a pas non plus de moyens humains nouveau. Il n'y a pas de d'inspecteurs en plus dans les inspecte dans dans les instituts régionaux de formation, donc voilà, la question des moyens, elle est posée, on crée des choses. Sans aucun moyen. Et comment voulez-vous avec ça : assurer la qualité de l'enseignement, alors que c'est vraiment essentiel pour assurer la crédibilité et l'avenir de l'enseignement français à l'étranger sur la durée mais aussi le respect des familles qui mettent leurs enfants dans la maison.

qui est essentiel, qui est celui de la formation et de la formation, donc des enseignants et plus partie quand même ceux qui sont sous statut local, si je puis m'exprimer ainsi, essayer de faire de telle sorte que cela puisse répondre à des attentes qui sont les attentes des établissements et et c'est un élément important, cet homme, cet article aussi vise à à conseiller les les promoteurs d'initiatives en vue de la création d'établissements d'enseignement, et ça je crois que c'est un élément important comme celui-là, linéaire, qui suit d'instruire les dossiers de demande de garantie de l'État pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement. Tous ces établissements du réseau de la EFE sont importantes pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger, mais sont aussi un outil important et essentiel de rayonnement de la France et de rayonnement de la francophonie dans nombre de ces pays j'ai en mémoire déplacement parlementaires que que j'avais fait, il y a, il y a, il y a quelques années, dans un pays d'Amérique centrale, qui par définition n'était pas francophone et tous les entretiens que nous avons eue avec les ministres membres du gouvernement de ce pays se sente tenus en français essayant de comprendre pourquoi cela en fait, ils étaient tous passés par le lycée français du pays concerné, et cela finalement nous montrer que étonnant, un outil tout à fait intéressante de rayonnement donc dans notre pays, j'allais dire de stratégie d'influence à à certains égards, et à l'heure où nombre de pays essaye de développer des réseaux d'influence, nous nous avons une chance extraordinaire inestimable, par le biais de ces réseaux et donc au travers de ce texte de loi, nous allons lui donner encore plus de moyens pour pouvoir prospérer et c'est un élément important et essentiel.

on attend en effet de la loi que dans 2 articles successifs l'expression utilisée soit identique et donc on comprend que l'article 3 listes, les missions de l'agence et l'article IV s'attache plutôt aux IRF mais nous pensons qu'il qu'il est nécessaire qu'il y a cohérence dans le texte, merci monsieur le président. commissions, sur cet amendement, de cohérence, le 12. Alors l'article 3 complètent la liste des missions confiées à l'agence en application du principe de spécialité des établissements publics, mais il n'a pas vocation à hiérarchiser ses missions alors j'avais une autre solution, madame. Madame Conway Mouret ne n'en veut pas, j'avais prévu, enfin, la commission avait prévu d'être d'accord avec l'amendement numéro 16 qui est à l'article 4 mais qui dit à peu près à peu près la même chose et pour être en cohérence avec le gouvernement, je donnerai donc un avis défavorable au 16 est favorable à ce que, au 12 qu'on discute actuellement voilà favorable.

Oui, monsieur le président je rappelle juste la vocation de la EFE et de former justement les personnels exerçant dans les établissements français de l'étranger dans le cadre de la formation continue en voulant élargir le public ciblé par les formations des instituts de régionaux de formation à des personnes ayant vocation à exercer dans les établissements français cet article ouvre une brèche qui pourrait nuire à l'opérateur public tout d'abord cette extension du périmètre de formation risque de s'effectuer au détriment de la formation continue des personnels des établissements français à l'étranger, on peut d'ailleurs s'interroger sur les critères de sélection de ces personnes ayant vocation à exercer et les garanties qui seront mises en place pour s'assurer qu'elles exercent bien in fine dans les établissements français de l'étranger, ensuite, on peut se demander s'il est normal qu'il revienne au contribuable français de financer la formation de personnes qui pourraient ne pas enseigner dans le réseau de la AFE donc on on souhaite apporter une vigilance pour que RF finalement ne soit pas dévoyé et détourné en un outil de privatisation des engagements supplémentaires de la part de de l'État français, donc, cet amendement, il a, il a donc pour objet de limiter les formations proposées par les IRF à la formation continue des personnels déjà recruté tels que veut la mission de la EFE afin d'éviter jusque IRF ne favorise la création d'établissements concurrents aux établissements homologués du réseau. Sous le président Monsieur le ministre, les IRF doivent assurer la formation de professeur, déjà présente dans le réseau, ainsi que celles de personnes ayant je cite vocation, il y a exercé l'ouverture de l'information à cette catégorie de personnes, pose de nombreux problèmes : celui de la sélection de ces personnes du diplôme qu'ils obtiendront et de la possibilité qu'elles viennent enseigner en France alors qu'elles n'ont pas passé du concours ou bien encore le fait qu'elle concerne bel et bien, à l'issue de leur formation dans une école française à l'étranger, trouvez-vous normal que des instituts subventionné par la France forme des personnels qui pourront exercer dans les systèmes éducatifs étrangers ou bien encore que ces personnels uniquement formé au sein de l'IRF puissent, au même titre que nos professeurs enseigner dans nos établissements, que cela soit en France ou à l'étranger, ma crainte est que l'on crée ainsi une nouvelle catégorie de personnel et qui, à terme, vient de remplacer les titulaires de l'Éducation nationale, au sein des établissements d'enseignement français installés à l'étranger, or ce sont bien eux qui sont les garants de la qualité pédagogique de nos lycées, la formation continue des personnels français est ainsi un exemple, la création des IRF assurant à la fois la formation du personnel du réseau et la formation de futurs personnel risque d'entraîner des difficultés d'accès et un appauvrissement des cursus destiné au personnel déjà en place, donc, cet amendement vise à demander la suppression de l'expression ayant vocation à. mais non. Alors là, la question qui est posée est importante et structurante dans la réforme, c'est l'un des points centraux de cette proposition de loi, en effet, l'avait fait, se voit confier par cette proposition de loi, une mission de formation qui va bien au-delà de la seule formation continue de ces personnels, les instituts régionaux de formation sera en effet habilité à former, non seulement les personnels du réseau. Mais aussi les personnels ayant vocation à exercer au sein de et des personnels des systèmes éducatifs étrangers au titre et c'est important, au titre de la coopération éducative, le ministère de l'Éducation nationale promet 1000 détachement, comme je le disais tout à l'heure d'ici à 2030, mais ce ne sera pas suffisant pour soutenir la croissance du réseau, il s'agit donc ici de créer des cursus diplômant qui garantiront l'existence d'un vivier de personnel disposant d'un niveau de qualification conforme aux exigences de qualité des enseignements et aux critères de l'homologation ces cursus sont déjà expérimentée dans certains réseaux ayant des besoins importants ou en développement au Maroc Liban en Égypte, il fonctionne sur la base d'un partenariat entre une institution d'enseignement supérieur, lequel Institut national supérieure du professorat et de l'éducation français la la forte croissance prévisible du personnel de droit local appelle l'extension de ce type de dispositif et je vous proposerai toutefois d'adopter à l'article IV non mais je vous pose on on ne pas parce que je viens de dire que non, donc l'avis est défavorable.

ils viennent de défendre devant vous l'entrée des dispositifs flamme au conseil d'administration pour nommer que celui-ci de l'agence d'enseignement français à l'étranger et là dans ce que vous dites en fait, vous êtes, vous de nous dire que vous voulez réduire au seul périmètre des établissements homologués alors que juste avant vous, de vous voulez donner plus de pouvoir finalement au dispositif flamme en interdisant à ses professeurs de venir se former dans ces instituts, pour moi, il y a une forme de d'incohérence complète, hein, mais peut-être que vous précisera après donc pour pourquoi il me semble assez. Je je dirais a assez peu, je dirais, là pour le coup, bienvenue je de fermer à ce point saisi RFC c'est parce que tout simplement, aujourd'hui, nous en avons un besoin criant quand je vous dis, criant c'est que oui, nous avons besoin à la fois qu'il puisse former un certain nombre de personnels en formation et je le redis et je l'assume pleinement initial dès lors où c'est nécessaire continue et de qualité pour l'ensemble des personnels du réseau, sans cela, effectivement, notre réseau finira par s'éteindre au bénéfice au bénéfice du modèle anglo-saxon, qui lui ne se pose pas ce genre de question donc je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment prendre conscience que c'est une chance extraordinaire que l'on offre à ce réseau, aux parents et surtout à nous-mêmes, de rester crédibles, crédibles dans notre enseignement français à l'étranger qui fait notre renommée, on ne peut pas aujourd'hui dire, simplement parce que nous défendons une corporation réduire à cette corporation dont j'ai fait partie. Et bien que on leur laisse simplement eux accès à la formation continue, non la formation initiale est nécessaire, moi j'ai été enseignante j'ai commencé ma formation initiale en France, il y en a bien voulu aussi avoir cette formation initiale à l'étranger, pardon, je suis passionné mais moi ce réseau, c'est ma vie et quand j'entends certaines choses, je me dis qu'il faut rectifier certaines choses. Madame, chers collègues, quels que soient vos états d'âme, le temps de parole et le temps de parole et vous le respecter comme tout le monde ici et vous le respecter, sinon je le ferai respecter et je serai dans l'obligation de le plus vous donner la parole. Merci.

celle des recrutés locaux, compte tenu du poids croissant dans les effets qui du réseau depuis 2017, 2 ceci, puisque, en effet, leur nombre a augmenté de 9 % mais en fait, ce qui pose problème c'est la rédaction actuelle des articles 3 et 4 qui soulève un grand nombre de questions quant à la vocation des instituts régionaux de former les personnels ayant vocation à exercer dans les établissements français à l'étranger ces questions, a déjà été posée par les orateurs précédents mais on se demande, en fait, ce que cette expression cash ou comprend les contours en sont très flous et quand c'est flou, vous savez, voilà où donc ouvre-t-elle la formation à des personnes qui ne sont pas des enseignants, quels sont les critères qui seront choisis cette formation débouchera-t-elle sur une certification et, le cas échéant, laquelle voire diplômante en fait c'est ce manque de clarté qui nous pousse à proposer la limitation des formations dispensées par les instituts régionaux de formation personnels exerçant effectivement dans le réseau. Merci, Monsieur le Si Monsieur le Président, ces milices, mes chers collègues, chers collègues, Samantha Cazebonne ce que vous décrivez, c'est tout le problème de l'éducation nationale qui n'arrivent pas à recruter suffisamment d'enseignants. En France, et aussi à l'étranger, donc effectivement se trouver des solutions et ça peut en être une, toutefois, je ne crois pas, non plus, que ce soit une baguette magique, dans la mesure où, comment voulez-vous trouver est ce que vous pensez vraiment. Que d'un seul coup de rien on peut arriver à quelque chose qui résoudra tous nos problèmes de, de, de, de, de on n'aura pas plus d'un inspecteur, par un un, un par un institut de de de régional de formation et que ses inspecteurs passe aujourd'hui plus de 60 % de leur temps à homologuer de nouveaux établissements pour dire regardez s'accroît. Donc, ils ne pourront même pas exercer leur leur leur fonction, ils n'exercent plus leur fonction dans les établissements, ils ne pourront pas exercer leur fonction dans les instituts régionaux de formation parce qu'il faut continuer à homologuer des établissements pour dire : regardez, on est en train de, de respecter les objectifs du président de la République, donc je ne pense pas qu'il faille penser que c'est une baguette magique, c'est utile mais c'est pas la solution absolue et deuxièmement, même si je reconnais que ce que vous nous indiquez sur flamme établi les peut nous mettre un peu en contradiction sur le fond, ce que nous disons ce que nous disons c'est : premières commençons déjà commençons déjà par le fer avec les personnes qui sont déjà dans notre réseau, il y a déjà un besoin sérieux, commençons par cela et nous verrons ensuite et d'ailleurs je ne sais pas si je ne sais pas, d'ailleurs, si quelque chose de plus est envisagée dans la mesure où il y a déjà une note hein de la greffe du du 9 décembre dernier qui a été présenté à son c'était qui indique très clairement les missions et attributions des instituts régionaux de formation donc avant même la discussion de cette PPL et qui n'envisage absolument pas cette ouverture à des personnes qui ne sont pas encore dans le réseau, et si c'était le cas, je crois que ça poserait en plus d'autres difficultés parce que nous créerons des établissements d'enseignement supérieur, d'une certaine manière, dans différents pays sans avoir discuté de leur statut et je crois que ça c'est quelque chose qui n'a pas encore été abordée dans le débat et qui pourrait être une difficulté complémentaires donc commençons déjà par faire ce dont nous avons besoin et dont nous savons que nous pouvons le réussir. Oui merci monsieur le président, moi j'entends les les inquiétudes donc qui sont formulées par ceux qui redoutent la concurrence des établissements étrangers qui, à les entendre, profiteraient de l'aubaine pour former leurs enseignants sur le dos du contribuable français, mais cette formulation est indispensable parce que, justement, ces nouveaux enseignants sont nécessaires, on a besoin de former des nouveaux enseignants pour accompagner le développement du réseau, c'est nécessaire, donc ils n'ont pas encore enseigner dans le réseau, mais ils vont, ils à enseigner dans notre réseau des écoles françaises à l'étranger, mais il y a besoin de mettre aussi cette vocation est d'ouvrir parce qu'on a un autre système qu'on cherche à développer et qu'on développe toujours avec la EFE c'est le Label France Éducation donc on pourrait très bien effectivement avoir des enseignants qui virait et enseigner dans un établissement étranger mais dans le cas du Label France éducation, ça pourrait être ouvert grâce à ça, donc je pense qu'il faut se préserver cette ouverture qui est nécessaire pour accompagner le développement du réseau, et encore une fois, chaque fois, vous mettez des limites, vous envoyez des enfants vers les systèmes étrangers. Merci, je vais mettre aux voix les amendements identiques 11 et 24 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Ils sont rejetés, 3 amendements en discussion commune le 26 Madame Garabédian. monsieur le ministre, en continuité dont présentant abondement, nous sommes tous très attachés à la francophonie, mais est-il juste que la France finance des formations de personnel, a priori, de nationalité étrangère qui exercent dans des systèmes étrangers : le coût de la création de six IRF et de leur fonctionnement n'est en effet n'est pas neutre pour les finances publiques, même si aujourd'hui c'est pas chiffré le bénéfice des formations devraient donc exclusivement être réservé au personnel d'établissements du réseau mon amendement vise à demander la suppression de cette formation aux personnels exerçant dans le système éducatif étrangers. il s'agit de répondre à l'objection légitime formulées par l'amendement numéro 13 de Madame tout en préservant la portée de la disposition par la commission, qui précise que les formations dispensées par les instituts régionaux de formation sont francophones, ces formations doivent avoir lieu en français si l'on souhaite que les instituts régionaux de formation contribue réellement à notre diplomatie culturelle des influences, c'est-à-dire que la UFE reste dans son rôle, cette disposition nous a paru d'autant plus nécessaire que ces formations seront ouvertes à un large public, nous avons eu l'occasion d'en débattre et la greffe n'aurait pas vocation, par exemple à dispenser des formations en anglais à des personnes ayant vocation à exercer dans le réseau ou exerçant dans des systèmes éducatifs étrangers qui pourraient décider ensuite de rejoindre le réseau anglophone, l'ajout de l'adverbe principalement qui ressemble beaucoup à notamment, j'en conviens, vide en fait de sa portée la disposition introduite par la commission, ils sont toutefois qu'une souplesse soit nécessaire dans certains cas précis et limités, c'est pourquoi je vous propose cet autre amendement prévoyant la possibilité d'exception dument motivée. Le 13 mai Derek Conway Mouret, même si vous avez déjà la réponse, mais bon. je, je pense que la la la rédaction du texte risquerait de priver certains personnels de de formation pédagogique, c'est-à-dire technique et je pense par exemple à certains personnels administratifs essentiels au fonctionnement de nos établissements, mais aussi à des professeurs de langues étrangères, qui sont des locuteurs natifs et dont le français n'est pas la langue maternelle, donc cela reviendrait finalement à exclure ces personnels-là et je pense que dans un souci de précision notre amendement propose donc de laisser ouverte la possibilité à la greffe de dispenser des formations pédagogique en langues étrangères, quand cela est nécessaire, ça peut être aussi la langue locale. Alors sur le 26 il s'agit de supprimer la possibilité pour le FE de former des personnels de système éducatif étranger au Tir de la ration éducative cette coopération éducative figurent parmi les missions assignées à l'avait fait depuis sa création, les auteurs de l'amendement parle d'ingérence, je parlerais plutôt d'influence mais aussi et surtout de contribution à la consolidation du système éducatif dans des pays disposant de compétences et de moyens insuffisants alors que l'éducation. Et l'acte est l'une des clés du développement, et s'il faut faire de la formation des personnels de l'AFP, une priorité, ce sur quoi nous aurons l'occasion de revenir plus tard, je vous propose de maintenir la possibilité d'actions de coopération éducative, donc l'avis est défavorable sur cet amendement numéro 26 sur l'amendement numéro 13 l'ajout du de l'adverbe principalement qui ressemblent beaucoup à notamment vite de sa portée la disposition introduite par la commission, c'est pourquoi je vous propose une autre formulation dans l'amendement que j'ai des des proposé de nature à satisfaire les auteurs de cet amendement, donc je lui demande, pour le 13 demande de retrait sinon avis défavorable. Avis du gouvernement sur les trois amendements. Merci Monsieur le Président, écoutez sur le 26 non, c'est un avis défavorable, c'est au coeur du rayonnement justement de de la langue française, le fait que de pouvoir travailler sur cette coopération

ça serait plutôt à l'Académie française, d'être l'arbitre des élégances, mais faute d'avoir ces qualifications moi j'avoue que j'ai une préférence pour le 13 parce que le 36 ils cadenassent beaucoup je trouve, et là aussi je sais pas, franchement, je suis un passionné de francophonie biberonné par le président Jacques Legendre ici donc voilà pour prendre des références, mais je pense que ce le le numéro 13 voilà donne plus de latitude pour aussi s'adapter à des publics en langue nationale et et faire en sorte qu'on partage tout cela, donc ce serait un avis défavorable, monsieur rapporteur au 36 et un avis favorable au 13 ans. Très bien. Madame, non, j'avais d'abord pardon, il y avait d'abord Madame Conway Mouret. Non. si vous y renoncer, c'est bien. elles sont quand même susceptible d'être assez nombreuses et si à chaque fois, elle demande l'instruction d'une demande, on peut imaginer que cela induira des formalités administratives supplémentaires, ce qui semble absolument pas nécessaire puisque la demande devra être dument motivés, donc qui en décidera, devra-t-on installer un comité pour les accepter et donc je pense que la rédaction que nous proposons à l'amendement, hé bien, répond au cas par cas en laissant une grande flexibilité, notamment pour la diversité des formations qui vont être proposés. Si Madame Cazebonne. je comprends enfin et vous avez raison, je partage avec vous l'envie de défendre au-delà tout la la francophonie mais il y a quand même un principe de réalité nos établissements France français à l'étranger, fonctionne dans le cadre d'accords bilatéraux, nous vivons dans des pays qui nous accueille, et avec lequel nous avons des conventions, je vous donne le cas que j'ai vécu, à savoir un lycée en Espagne où on enseigne dans le cas des accords, le Catalan,

et pour nommer que lui, hein, parce que je vous donnerai un autre exemple, derrière, il faut bien que je puisse le formé à la pédagogie française, donc ça veut dire qu'on va au moins lui parler dans la langue de transmission puisqu'on a des inspecteurs et contrairement à ce que disait monsieur le on a beaucoup plus que ce qu'il ne décrit, qui ont aussi cette capacité à enseigner dans plusieurs langues, mais c'est aussi le principe de notre réseau et donc quand c'est nécessaire dans. Dans la langue du pays puisque, sinon, nous n'avons pas de professeur, mais nous ne, surtout, nous ne pouvons pas répondre à la commande des accords bilatéraux dans lesquelles nous sommes engagés, voilà donc je rappeler quand même ce principe de réalité, parce que vraiment c'est celui dans lequel nous vivons et deuxièmement quand nous demandons à nos. Professeur de ce certifiés dans l'enseignement d'une langue par exemple enseigner les mathématiques en anglais, et que c'est un professeur français,

Très bien, allez je vais mettre aux voix, donc d'abord le 26 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté, le 36 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. 36 de la commission, je dis bien. Merci qui est contre. Il est adopté, il fait tomber évidemment l'amendement de presse. Le 32 madame Vogel. Oui, merci Monsieur le Président, très rapidement, comme je sais que vous aimez ça cet amendement est très simple : il supprime le Conseil de la greffe au promoteur d'initiatives en vue de la création d'un établissement, simplement parce que nous craignons que le conseil à l'homologation d'un opérateur chargé de doubler le nombre d'élèves posent un questionnement quant à la neutralité du Conseil qui serait donnée et puisse risquer de faire baisser les exigences de qualité sur les établissements homologués. Merci, avis de la commission. cet amendement conteste le rôle de conseil de l'agence auprès des candidats le l'homologation l'homologation est accordée par le ministère de l'Éducation nationale, elle a testé, reconnaît que les établissements dispensent un enseignement conforme aux principes au programme et à l'organisation pédagogique du système éducatif français l'attribution de l'homologation s'effectuent en accord avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères afin d'accélérer la croissance de réseau, conformément aux objectifs qui lui ont été fixées, la greffe a d'ores et déjà renforcé son rôle dans l'accompagnement des projets d'homologation en créant un service d'appuyer le développement du réseau ce rôle de conseil est essentielle pour alimenter la dynamique actuelle des homologations depuis 2019 l'homologation des établissements, accompagnée par l'OFCE a permis de faire entrer 9000 nouveaux élèves dans le réseau, une cinquantaine d'établissements sont actuellement accompagné ce rôle doit être confortée en étant inscrit dans la loi et donc la commission a émis un avis défavorable. Gouvernement même avis je mais on voit le 32 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui compte moi. Le 2, madame Gréaume. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il nous semble important d'inscrire l'action des établissements du réseau EFE dans l'ensemble des outils d'influence français dans ce cadre, il nous paraît nécessaire que ce dernier s'attelle à développer une relation avec les acteurs culturels institutionnels et médiatiques locaux l'enjeu ici est double : 1er s'est une nouvelle fois de faciliter l'intégration des familles au sein de leur pays de résidence ainsi, cela peut être une bonne méthode, que de faire découvrir aux enfants et indirectement par an, les établissements culturels des pays dans lequel parfois ils viennent d'arriver à ce titre-le renforcement des enseignements culturels et artistiques s'attend 5 ans après l'année de parcours d'éducation artistique et culturelle constitue un levier très prometteur, le second comme je l'ai évoqué ces deux permettent de mieux faire connaître le réseau auprès des familles françaises, mais aussi des familles étrangères si notre objectif est bien de doubler le nombre d'élèves, d'ici 2030, il est nécessaire de renforcer la visibilité de l'AFE et de ces établissements, cette action de promotion et de valorisation, les établissements et le réseau en lien avec le ministère des Affaires étrangères, le fait déjà, ils sortent donc légitime que cela soit inscrit officiellement dans ses missions, cela pourrait être d'ailleurs être utile à l'avenir et notamment au moment de renégocier le contrat d'objectifs et de moyens du réseau merci. c'est une idée intéressante, bien entendu, mais qui figure déjà au 3ème mois de l'article L 452 tiré 2 du code de l'éducation qui dispose que la greffe a pour objet de contribuer au rayonnement de la langue et de la culture française, le texte proposé serait donc redondant avec ce troisièmement, par ailleurs, cette nouvelle mission : créer une confusion avec l'action des autres acteurs publics, les services culturels des ambassades, l'institut français etc et donc la commission a émis un avis défavorable Je mais on voit le 2 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté, le 14 Madame Conway Mouret. Oui, merci Monsieur le Président, l'avait fait, encouragent les démarches innovantes et des approches pluridisciplinaires d'ailleurs cela a été rappelé par l'auteur, Samantha Cazebonne dans la discussion générale, elle a ainsi organisé son 1er forum de l'innovation pédagogique à Prague les vingt-quatre 25 janvier 2020 et a réuni plus d'une centaine de participants afin de préparer l'école de demain et faire évoluer les pratiques depuis 2010, elle a aussi intensifié son par tonne Aria, je vais y arriver avec le CNED afin d'assurer la continuité de l'offre de scolarisation française dans tous les contextes et s'est avérée précieuse d'ailleurs pour traverser la crise sanitaire mondiale, donc il nous sommes important d'inscrire dans le code de l'éducation, le rôle de l'avait fait en tant que laboratoire d'innovation pédagogique, qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs fixés par le dernier contrat d'objectifs et de moyens

si l'enseignement des langues vivantes débute désormais à l'école élémentaire, les professeurs des écoles sont peu formés et souvent mal à l'aise. Avec cet enseignement, or dans ce domaine de l'apprentissage des langues, il y a beaucoup à prendre les systèmes scolaires étrangers et les établissements de la EFE peuvent servir de relais, l'agence développe des dispositifs d'excellence dans ce domaine, section européenne orientale et international des parcours renforcée en langues étrangères sont proposés dès le CP les élèves évoluant naturellement dans 2 langues, le français est la langue du pays, d'autres l'idée de que cette expérience puisse être source d'enseignements pour l'éducation nationale est intéressantes et même pertinentes et donc la commission a émis un avis favorable, Donc. Ce sera une sagesse. Ben voilà Madame Conway Mouret, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, allez donc sur le 14, j'ai un avis favorable de la commission sagesse du gouvernement qui est pour.

qui est contre qui s'abstient, il est adopté. à l'article IV 4 amendements en discussion commune le 33 madame Vogel. Oui, donc, cet amendement propose de modifier la rédaction à la fin de l'alinéa qui parle de la du fait que la formation continue de personnel et prioritairement fait fait pour les personnels qui ont vocation à travailler dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, donc le but de l'amendement c'est de clarifier que la mission principale des IRF c'est la formation continue des personnels du réseau, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire que ça, qui doit faire que ça, mais ce que c'est, mission principale ou de personnel qui exerceront effectivement dans le réseau, donc on a mis sous réserve d'une promesse unilatérale de contrat parce qu'on comprend bien que dès que 2 des personnels qui vont vraiment enseigner mais dont le contrat a pas encore commencé, peuvent tout à fait avoir vocation à être déjà formés et il précise : à la fin que l'on peut dans certains cas, assurer des missions de formation au bénéfice de personnes existe exerçant dans les systèmes éducatifs mais on a mis une procédure en disant que c'est dans certains cas, définis par l'agence après consultation de l'instance de gouvernance pédagogique et scientifique des IRF, ce qui permet, dont les détails seront précisés précisés par par voie réglementaire, mais qui permet disons de contrôler un peu la manière dont les formations pour du personnel au réseau serait faite. Merci le 16 Madame Conway Mouret. Oui, merci Monsieur le Président, bon, d'abord, cet amendement vise à garantir la cohérence du texte puisqu'il y a eu, il renvoie à l'amendement. En assurant le caractère prioritaire de la formation des personnels exerçant au sein de notre réseau à la fois donc aux articles III et IV cette priorisation nous sommes nécessaires pour plusieurs raisons : d'abord parce que la proposition de loi change substantiellement la mission qui incombe à la Uffe puisque jusqu'à présent, au titre de l'article L 452 du code de l'éducation, l'agence avait pour objet de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers, il était alors un partenaire des postes diplomatiques chargé de cette mission mais l'alinéa 7 de la proposition de loi ajoute que l'agence contribue à la formation de personnel exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers et donc elle devient le, l'acteur principal de cette mission de coopération, deuxièmement nous souhaitons cibler prioritairement les personnes exerçant au sein du réseau afin que ceux-ci soient assurés de bénéficier de formations qui leur sont nécessaires en cas de forte demande, ce n'est rien, exclusif, bien sûr, d'une demande locale des professeurs, employé au profit d'une formation initiale pour répondre aux besoins d'autres systèmes éducatifs, en fait, ce que nous proposons, c'est de gérer le développement des IRF éviter les tensions inutiles. Madame Renoux Garabédian, les 25 et 27 sont des amendements de coordination mais sur des amendements qui ont été rejetés, donc ils sont retirés les 2 merci. Commission donc sur les 33 F 16. concernant l'amendement numéro 33 rectifié, parce que je ne parlons pas des autres, l'amendement 33 rectifié, fait de la formation des personnels, une priorité tout en permettant au personnel qui serait sur le point d'exercer dans le réseau d'être formé en limitant les possibilités en matière de coopération éducative, les amendements 25 27 on ne discutera pas

Merci président avis défavorable sur le 33 rectifié et sur le 16, bon, on a déjà précisé une première fois, c'est vrai que le préciser une seconde fois peut être superflu, je me range à la sagesse de l'Assemblée. Madame Conway Mouret les retirer. Oui mais Monsieur le Président, c'était simplement pour la cohérence du texte c'est tout si on on affirme quelque chose dans l'article 3 alors qu'on fait la liste des missions, on réaffirme la même chose dans l'article IV c'était voilà

Qui est contre. Le 33 est rejeté, alors le 16 qui effectivement et avait elle-même texte que le 13 à l'article 3 mais bon ça ne change pas grand chose sur le fond, mais la vie est négatif sur la forme, pourquoi le redire alors qu'on a déjà dit, donc pour le moment j'ai un avis négatif, en tout cas de la commission pardon et sagesse du gouvernement qui est pour. Je suis rentré dans le vote, là Monsieur le comte, c'est un peu compliqué non. Donc, il est pour. il est pour. Il est rejeté, mais sincèrement, ça ne change pas grand chose, il est déjà dans l'article 3. 3. Oui, aussi, avec ça, qui n'étaient pas conformes au code de l'éducation. Allez l'amendement 28 Madame Renaud Garabédian. la gouvernance des IUFM est assurée par une instance administrative et financière d'une part, et par une instance pédagogique et scientifique, d'autre part, propre à chacune des zones, cet amendement vise à assurer la participation de représentants des enseignants aux instances pédagogique et scientifique. Commission. l'institut régional de formation et d'une interface qui assurera la gestion administrative et financière de l'ensemble des moyens déconcentrés de l'agence mutualiser l'échelle d'une zone géographique, ces moyens proviendront des contributions des établissements, c'est-à-dire d'une part, de la participation des établissements partenaires aux frais du réseau et d'autre part, la participation à hauteur de 1 % de la masse salariale de tous les établissements homologués pour financer les actions de formation, d'après les informations qui nous ont été fournis pour assurer leur mission les IRF seront donc doté d'un conseil des affaires administratives et financières regroupant des personnels de l'institut régional de formation et de l'agence des représentants des parents d'élèves et des personnels et des comités de gestion des établissements une seconde instance le conseil pédagogique et scientifique apportera l'expertise nécessaires pour l'élaboration d'un plan régional de formation et l'évaluation des actions menées, il est évident évidemment légitime que les enseignants participent à cette instance pédagogique et scientifique : avis favorable Merci monsieur le président, alors en fait, dans, dans, dans la gouvernance des désirs rêves les représentants des personnels, ils sont bien présents dans ce conseil des affaires administratives et financières et ce conseil, justement, il étudie il amende il valide le plan régional de formation et toutes les actions menées par les rêves, donc il nous semble que l'esprit et l'intention qui guide les eaux, l'auteur de l'amendement est satisfait par le dispositif mis en place le CPAS. En revanche, dans lequel il il souhaite intégrer ces ces enseignants n'est pas une instance d'identification des besoins c'est une instance d'ingénierie et donc voilà, nous, nous souhaitons rester au texte sorti de la commission avis défavorable. Le 28 à l'heure, amendement avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. j'ai dit favorable de la commission ah ben voilà, non mais vous n'écoutez pas, je me disais aussi c'est curieux, vous savez ce que c'est, aujourd'hui, elle est très bien qu'il est d'accord, qui vote contre L'amendement est adopté je mais on voit l'article IV qui est pour. Qui est contre, il est adopté, après l'article 4 le 17 monsieur le comte.

qui sont faits de titulaires de l'Éducation nationale vers l'enseignement français à l'étranger, aujourd'hui, vous le savez, il y a 2 types de détachement pour les titulaires de l'Éducation nationale, il y a d'une part, des détachements de l'Éducation nationale vers l'avait fait pour les établissements qui sont en gestion directe et conventionné et des détachements Direct vers les établissements qui sont les établissements partenaires et les détachements Direct c'est l'éducation nationale qui opère directement les détachements vers les établissements, on doit constater qu'alors que l'avait gère ça ressource en essayant de l'économiser, puisqu'elle est rare, nous n'avons pas assez d'enseignants et l'avait fait, n'a pas les moyens de les rémunérer, toutefois il doit constater une anarchie absolue et totale. des détachements Direct vers les établissements partenaires parce qu'en réalité à la DGA chez l'éducation nationale, personne ne s'en occupe et on doit donc constater qu'il y a une ressource qui est particulièrement mal répartis dans le monde, parce que finalement ça ne dépend que des établissements partenaires de savoir comment et à qui parler, à l'éducation nationale pour avoir des détachements nous donnons donc par cet amendement, un rôle à l'agence pour détacher et assurer une répartition. Juste, efficace de l'ensemble des détachements qui sont opprimés par les titulaires de l'Éducation nationale à l'étranger, je rajoute que lorsque vous détacher une personne titulaire des questions nationales directement auprès d'un établissement partenaire, ça représente un coût caché d'à peu près 25 à 30000 euros par an en terme de pensions civiles, il s'agit donc finalement d'une dépense de l'État significative qui peut être justifiée mais qui mérite d'être également répartie et correctement, c'est l'objectif de cet amendement. Commission. Alors, la situation des personnels détachés par catégorie d'établissements est la suivante : premièrement, l'agence affecte des personnels titulaires expatrié ou résident détachés dans les établissements en gestion directe et conventionné du réseau, et deuxièmement, par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale peut détacher directement des personnels titulaires au sein des établissements partenaires ces fonctionnaires détachés sont alors recrutés dans le cadre d'un contrat de droit local 1000 détachements supplémentaires de personnes titulaires de l'Éducation nationale ont été promis à l'horizon 2030, ce qui pose en effet la question de la coordination dans quelle mesure l'EFE pourrait-elle assurer une fonction de coordination alors que ces détachements sont décidées par le ministère de l'Éducation nationale en fonction des besoins des établissements partenaires des besoins recensés en France. Dans les académies et des situations individuelles des fonctionnaires candidat au détachement les établissements partenaires sont-ils demandeurs d'une telle coordination, il s'agit en définitive de mieux coordonner les actions du ministère des Affaires étrangères du ministère de l'Éducation nationale dans le domaine de l'enseignement français à l'étranger, que proposez-vous en ce sens, monsieur le Ministre, la commission souhaiterait connaître l'avis du gouvernement. Non mais c'est quoi à votre avis. C'est quoi l'avis de la commission non mais l'avis du Gouvernement mais en fonction de l'avis du gouvernement, la commission s'aligne la commission s'aligne sur l'avis du gouvernement, d'accord, avis du Gouvernement. Merci monsieur le président, alors en fait je pense que la rédaction de l'amendement de de Monsieur, le comte n'est pas totalement en ligne avec l'exposé des motifs et ce qu'il vient de défendre je lis de L 452 5 du code de l'éducation, je l'ai sous les yeux, en réalité, l'amendement qui propose, hé bien, visent à une remise en cause significative des statuts existants, ça signifierait que les détaché auprès de la UFE ne serait plus auprès de la EFE mais auprès des établissements, ce qui signifie la disparition pure et simple des statuts d'ailleurs de résidents et d'expatriés, donc les détacher serait dès lors considérés comme des détaché Direct et recrutés sous contrat local par les établissements, ça c'est l'effet concret de l'amendement et je pense pas que Monsieur le comte, que ce soit l'effet recherché, de sa part, donc voilà, mais a donc un avis défavorable. Il est maintenu, monsieur Leconte attendez, attendez, on va voir si d'abord Monsieur le comte le maintien après les propos du ministre. Monsieur Leconte il est maintenu ou non.

j'ai eu le problème, c'est que j'ai, j'ai dû évoquer ce sujet par cette par ce biais d'amendements de coordination, alors que l'autre m'a été imposé, article 40, non, non, non, mais je, je reconnais, c'est pour ça que je me retire, je retire l'amendement. Et retiré mais c'est un sujet majeur sur lequel j'aurais entendu bien entendre le gouvernement parce que c'est majeur pour l'avenir de l'enseignement français à l'étranger si les retirer, il y a pas d'explication sur ce qui est retiré allez. Un amendement et un sous-amendement le vin monsieur Leconte. Merci de demander à d'un. Inscrire dans dans le code de l'éducation qui comprend déjà un rapport à l'Assemblée des Français de l'étranger, le fait que chaque année dans ce rapport, l'agence inscrits les futures évolutions des instructions des bourses scolaires et du barème de bourses scolaires de manière à ce que ça puisse être débattue au sein de de l'assemblée des des Français de l'étranger car il est important que cette cette cette politique des bourses scolaires fassent partie finalement des débats à l'Assemblée des Français de l'étranger, dans un cadre et avec des éléments qui sont. à chaque fois qu'il y a des modifications, il faut qu'elle puisse être débattue à l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est la raison pour laquelle nous proposons l'inscription de ce site dans le code de l'éducation. Merci le sous-amendement 38, monsieur le rapporteur. Alors ce sous-amendement propose d'insérer les informations demandées par l'amendement numéro 20 dans le rapport de l'AFP au Parlement plutôt que dans son rapport à l'Assemblée des Français de l'étranger, laquelle pourra néanmoins disposer ainsi également de ces informations. Monsieur le rapporteur, tant qu'à faire, donnez-moi votre avis sur l'amendement 20 j'imagine. La Commission partagent ce souci de transparence ne souhaiterait que ces informations soient portés à connaissance du Parlement, d'où le sous-amendement. Donc nous serons avis favorable, si le sous-amendement est voté. Très bien, avait du gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement. en réalité, ces informations sont communiquées lors de la commission nationale des bourses, des représentants de l'AFE sont à cette commission nationale des bourses à chaque fois l'AFE tous les sujets seront débattus, donc il n'y a pas d'obstacle à ce que ce sujet soit débattu à l'AFE, de façon générale et donc franchement je vois, je vois pas d'objets réels au regard de la pratique et dans les commissions nationales et au sein de l'AFE et donc c'est un avis qui était défavorable et à l'amendement et jusqu'à maintenant. monsieur le président, monsieur le rapporteur, en fait, l'idée d'abord. C'est le le rapport comprend l'ensemble des composantes du barème et les propositions d'évolution des instructions de la prochaine campagne de bourses scolaires il s'agit donc de permettre par mon amendement à ce que l'AMF présente d'inscrire dans la loi que l'AMF présente à l'Assemblée des Français de l'étranger, ces propositions d'évolution pour que la greffe en débattent et éventuellement émettre des remarques, ça n'est pas la même chose qu'un rapport a posteriori et donc nous nous je, je, je, je crains que si vous souhaitez simplement une information du Parlement plutôt que permettre à l'AFM à l'Assemblée des Français de l'étranger d'en débattre, auparavant, que nous perdions finalement les. Prix de cet amendement, l'esprit de cet amendement, c'est de permettre à l'Assemblée des Français de l'étranger, de pouvoir débattre des évolutions futures du barème et donc je ne pense pas, monsieur le rapporteur, que votre amendement améliore les, les, les, les, les choses bien au contraire, parce que ce n'est pas au Parlement que nous débattrons du barème des bourses scolaires de la D. D. de par les la l'Assemblée des Français de l'étranger, la par la greffe, mais bien à l'AFP. Monsieur le comte, vous êtes bien conscient que si le sous-amendement est voté, mais que l'amendement ne l'est pas, tout tombe. je mais on voit donc le sous-amendement 38 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient. Il est adopté, je mets maintenant aux voix l'amendement 20. Avec un avis favorable de la commission puisque le sous-amendement est voté et un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Finalement, le vote. Qui est contre, il est adopté, donc adopter, sous-amendé, telle qu'indiquée, le 18 Madame Conway Mouret. Oui, au vu de du sort réservé à nos amendements qui qui tente d'état à apporter des des réponses au au blocage financier qui empêche à l'agence de se développer aujourd'hui, alors que par ailleurs elle doit procéder à la restauration mise aux normes de certains locaux ainsi que l'extension de son parc immobilier pour accueillir les nouveaux élèves ce que nous pensons, c'est que nous aurons peut-être la possibilité, par le biais d'un d'un rapport que le Parlement soit informé pour répondre, entre autres, aux interrogations des rapporteurs pour avis budgétaires qui chaque année font état des déblocages d'une agence qui a des objectifs qui lui sont demandés mais qui n'a pas forcément tous les moyens pour les remplir

ce qui se traduit par une augmentation importante et annuel des frais de scolarité qui permettent de financer des travaux qui bénéficieront seulement aux générations suivantes d'élèves avec les conséquences que l'on on connaît sur l'et sur les la seconde est de recourir aux avances de l'Agence France Trésor, théoriquement destiné à un besoin de financement imprévus donc inadapté au financement immobilier alors le comme en tout cas le dernier prévoit d'ailleurs leur extinction en 2022 ou en 2023 et le remplacement par un nouveau mécanisme. Qui au demeurant ne semble pas très adéquate et qui sera étudié par un groupe de travail interministériel, donc nous pensons que, que ce rapport bien permettrait peut-être d'avoir des réponses aux questions que nous nous posons depuis très longtemps à la commission des Affaires étrangères de la Défense et et des forces armées et d'essayer de remédier une fois pour toutes et trouver une solution pour essayer de débloquer, hé bien c'est à eux qu'il ne peut pas contracter d'emprunt supérieur à 12 mois. comme je l'ai déjà indiqué dans la discussion générale, la principale entrave au développement du réseau réside aujourd'hui dans l'interdiction faite à l'OFCE, d'emprunter à moyen et long terme alors que des opérations immobilières sont nécessaires pour accroître les capacités d'accueil des établissements en gestion directe, j'espère que nos débats d'aujourd'hui permettront des avancées sur cette question cruciale de l'endettement qui se négocient avec Bercy, c'est un point de blocage important sur lequel le Parlement ait empêché d'agir du fait de l'article 40 de la Constitution, il serait regrettable de devoir se passer de la contribution des hauts GD à la croissance du réseau, alors que votre ministère, l'ambition de doubler à terme les effectifs lors de la création de la il était prévu que celle-ci puisse emprunter cette disposition figure toujours l'article L 452 7 du code de l'éducation, mais elle a été abrogée, de façon implicite par la loi, comme je le disais, de 2011 et 2014 qui interdit aux organismes d'emprunter, nonobstant, donc je vous l'ai déjà dit, seule une loi financière pourrait revenir sur ce dispositif est encore faudrait-il pour que ce soit recevable, que ce soit à l'initiative du gouvernement une solution plus simple consisterait à ne pas classer la EFE comme ODAX ça a été proposé, il existe 700 soldats que je l'ai déjà dit leur liste est établie par l'Insee est fixée par arrêté du ministre de l'action des comptes et des j'ai évoqué de piste, il en existe peut-être d'autres, toujours est-il, Monsieur le Ministre, qu'il faut trouver une solution, le rapport proposé par cet amendement est donc le bienvenu, l'avis est donc favorable. Sur le rapport avis favorable de la commission. Favori. On aura tout vu le gouvernement. Il me semble que le Sénat avait un goût immodéré pour les rapports n'avait, parce que c'est pour étayer mon argumentation président dont vous voyez où je veux en venir dans dans dans la position du gouvernement, c'est que nous sommes désormais dans l'action, on n'est pas dans la compilation de rapports, on est dans l'action, on a un dispositif alternatif, les textes ont été pris une commission interministérielle va se réunir pour statuer sur les, les, les demandes d'établissements qui ont besoin de prêts garantis par l'État, donc voilà Action feu, on y va, pas besoin de rapport avis défavorable. Allez je mais aux voix l'amendement 18 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Merci qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Madame Conway Mouret un autre rapport le 19. Pardon, monsieur le président, oui, l'examen de cette proposition de loi nous permet d'évoquer largement les missions qui incombent à la UFE que l'article que 3 complète l'une d'elles, inscrite dans le code de l'éducation et de contribuer au rayonnement de la culture française dans les principes républicains et en particulier le principe de laïcité sont structurants, alors que le plan de développement de l'enseignement français à l'étranger, présenté en octobre 2019 a allégé les critères d'homologation afin de faciliter la création de nouveaux établissements, nous sommes plus que nécessaire de nous assurer du respect des principes cardinaux de l'enseignement français tels que l'égalité des chances et l'égalité entre les filles et les garçons dans l'ensemble du réseau, c'est la raison pour laquelle notre amendement demande au gouvernement un rapport qui nous permettrait d'avoir une vision globale des situations très diverses, qui peuvent exister au sein de nos établissements à l'étranger, alors bien sûr, monsieur le ministre, vous, vous avez cette vision-là, mais l'idée d'avoir un rapport c'est de pouvoir la partager avec avec le Parlement, ce rapport en dressant un état des lieux pourrait également permettre aux instituts régionaux de formation, de mettre en place des soutiens spécifiques à destination des personnels qui en auraient besoin, comme. Cela est le cas aujourd'hui dans l'Hexagone, voilà donc c'est un rapport qui permet à la fois de voir l'évolution du du réseau et puis de nous donner au Parlement, une vision de de celle-ci. l'homologation d'un établissement en tant qu'établissement français à l'étranger, attestent normalement du respect des principes, des programmes et de l'organisation pédagogique du système éducatif français mais nos principes républicains et en particulier le concept français de laïcité sont souvent mal compris à l'étranger, un état des lieux sur cette question paraît donc fort utile et la vie est favorable. Elle est vie du gouvernement, je préfère ne rien dire, monsieur le rapporteur. Eh bien, vous voyez, Monsieur le Président, au risque de vous surprendre, ce sera un avis favorable également parce que il y a tellement à mettre en valeur de ce qu'il est conduit par l'enseignement français à l'étranger, mise en place d'un réseau de ça ce correspondants laïcité mise en place d'une équipe, valeurs de la République pour l'UFE, bref, donc c'est un rapport qui est bienvenu : avis favorable. Les jeux mais au voile 19 avec 2 avis favorable qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Le 34 madame Vogel. Merci monsieur le président, donc c'est encore un amendement qui demande un rapport, cette fois-ci, un rapport sur l'état de la mixité sociale dans le réseau, nous l'avons dit dans un contexte où nous avons un désengagement de l'État, une réduction des bourses et bien les frais de scolarité augmentent et il y a un risque que la mixité sociale à l'intérieur du réseau France d'enseignement français à l'étranger, diminue et nous pensons qu'il serait utile pour pouvoir être mieux guidés sur le développement du réseau et les politiques publiques à mener dans le futur, de pouvoir se baser sur des données précises en ce qui concerne la mixité sociale et son évolution à savoir est ce qu'elle est maintenue, est ce qu'elle diminue et c'est pour cela que nous avons donc proposé cet amendement, je vous remercie. Sous-amendement 37 de la commission. Sous-amendement 37 de la commission. ils n'ont souvent pas choisi leur affectation et exerce une mission au service de l'État, l'existence d'un enseignement français à un coût abordable permet bien souvent d'éviter l'éclatement des familles et de garantir des affectations plus pérenne, mais le coup des établissements français à l'étranger est très variable et parfois très élevés dans ce contexte, les aides à majoration proposés sont-elles toujours suffisante et adaptée aux évolutions parfois rapide des frais de scolarité ce sous-amendement propose que le rapport proposait à l'amendement 30 34 soit aussi l'occasion de faire un point sur cette question. ben d'abord, la Commission va me donner son avis sur le 34 mais j'imagine que si elle le sous-amende, ce qu'elle y est favorable. Tout à fait, monsieur le président. Et le gouvernement sur les 2. aussi le gouvernement, il a été dans l'action, président on a assoupli la quotité exigibles 21000 à 23000 euros, on a mis en place plus de bourse 95 Meuros plus 13 ça fait 108 contre donc ça c'est pour démonter quand même des, des, des, des fausses informations qui ont été relayés à la tribune, précédemment, mais voilà sagesse si tout cela peut se traduire, noir sur blanc, voilà sa gestion. Sur les 2 sur les 2. Bon alors je mais on voit d'abord le sous-amendement 37 de la commission avec un avis de sagesse du gouvernement qui est pour.

Qui est contre, adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi est ce qu'il y a des explications de vote monsieur Leconte naturellement Madame Cazebonne madame Gréaume le elle doit maintenant hein, ne me faites pas le. Pardon, Oui, le prix, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voterons pour cette proposition de loi, dans la mesure où effectivement la porte sur un certain nombre de points des des éléments utiles à l'évolution de l'enseignement français à l'étranger nous émettrons aussi par cette explication de vote un certain nombre de réserves, car nous sommes pour la croissance du réseau, mais pour une croissance raisonnée, une croissance qui maintient la qualité, une croissance qui permet le développement et l'approfondissement des valeurs de l'enseignement français à l'étranger, nous ne sommes pas pour un grand bond en avant, une politique du chiffre. Il est important que, surtout dans un moment où, en plus, l'enseignement français évolue, il y a une place du contrôle continu, qui est plus importante que les questions, la question de l'homologation mérite un un suivi très au moment de l'attribution de l'homologation mais aussi par la suite, nous pensons qu'aujourd'hui. Pour garantir la qualité de l'enseignement français à l'étranger, nous n'avons pas les moyens de permettre cette croissance telle que voulue par le gouvernement, donc nous voterons pour cette proposition de, de, de, constatons que de la part du gouvernement, nous n'avons pas obtenu de d'assurance sur des moyens permettent. Temps de maintenir la qualité d'enseignement dans, dans, dans le cas de cette croissance du réseau, alors que la qualité, c'est ce qu'il y a de plus précieux : l'image de marque de notre de notre réseau, c'est le fruit de la mobilisation de tous les acteurs depuis des dizaines d'années. Et pour le maintenir et et le renforcer, nous ne pouvons pas aller dans une marche en avant vers la croissance sans maintenir la qualité. Et nous avons donc besoin de d'assurance sur des moyens aujourd'hui, nous ne les avons pas et nous n'avons pas non plus voté monsieur le rapporteur suffisant de les garanties que nous proposions pour assurer que les évolutions soient effectivement faites dans un cadre où la croissance du réseau s'accompagnent d'un maintien dans tous les cas de, de, de la qualité de l'enseignement, donc nous méritons favorablement, mais avec un salaire de. Monsieur le comte avant de donner la parole à Madame Cazebonne, je précise tout de suite que j'ai une demande de scrutin public par le groupe RDPI sur l'ensemble du texte, merci de vous y préparer Madame Cazebonne. Oui, merci, alors je je tiens tout d'abord à à remercier l'ensemble des groupes qui ont donné un avis favorable à ce à ce texte parce qu'il est fondamental, essentiel pour le réseau d'enseignement français à l'étranger, comme je le disais tout à l'heure, il est essentiel pour nos élèves, avant tout, bien sûr, pour les familles, on en a beaucoup parlé, bien sûr, pour les enseignants, on en a aussi beaucoup parlé, mais surtout pour l'avenir de notre réseau et et je tiens à rassurer le le sénateur Leconte sur le gage de qualité, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour la garantir cette qualité. Et je crois que, au moins, nous avons le mérite ensemble et je dis bien ensemble, hé bien d'offrir à ce réseau, l'opportunité justement de se qualifier encore plus qu'il n'a été puisque saisie RF. N'existait pas auparavant, désormais ils existeront et ils permettront. Comme nous le souhaitons tous, hé bien de faire de nos élèves toujours ceux qui sont reconnues pour leur excellence à travers le monde merci. Merci madame Gréaume. Malgré les limites que j'ai évoquées dans mon intervention générale notre groupe votera ce texte qui apporte quelques avancées au fonctionnement de la EFE toutefois il me semble que nous nous sommes face à une proposition de loi qui reste à l'écume des choses et que nous devrons nous à réinterroger sur l'ambition que nous avons pour le réseau et les moyens que nous sommes prêts à y consacrer, de fait, nous avons un équilibre subtil à trouver, d'un côté, il me semble que la UFE devrait permettre d'offrir un service public de l'éducation à l'ensemble des enfants de familles françaises expatriées de l'autre le réseau doit aussi permettent de participer pleinement à la scolarisation des enfants étrangers, notamment dans les zones géographiques où l'état des services publics et désastreux, car si la EFE ne fait pas, à proprement parler des opérateurs de l'aide publique au développement, il peut y contribuer fortement de par son domaine d'action son expérience au déploiement et son expertise à ce titre, et alors qu'on commence à peine à mesurer l'ampleur du désastre qu'a été l'option militaire au Sahel et malgré la montée en puissance de l'aide publique au développement, un renforcement de notre réseau éducatif et culturel à l'étranger est nécessaire au vu de cet objectif, la proposition de loi est clairement sous-dimensionné, on apprécie l'augmentation de la place des familles dans la gouvernance alors qu'elle finance la majeure partie du réseau mais c'est même ce modèle qu'il faudrait interroger pour justement démocratiser l'accès au réseau EFE et en faire un outil de rayonnement et de diffusion du modèle éducatif français je suis d'ailleurs assez sceptique et j'en terminerai par là par la volonté d'afficher de ne pas renforcer la logique partenariale entre la UFE et les systèmes éducatifs étrangers en atteste les débats que nous avons eue sur le périmètre des instituts régionaux, une formation, volonté d'aller plus loin que nous voterons ce texte merci. Merci avant le président Alizard quelques mois Monsieur. Merci monsieur le président, oui, pour conclure, c'est que quand on n'a pas la qualité, chers collègues, on ne peut pas faire croître un réseau donc forcément, si on veut le faire croître, on aura la qualité, et encore une fois s'opposer à la croissance du réseau c'est envoyé des dizaines de milliers d'enfants vers, justement des systèmes d'enseignement étrangers, donc si on veut effectivement accroître ce nombre d'enfants, il faut avoir cette dynamique, c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, dans les propos liminaire en discussion générale, le groupe centriste bien sûr va voter ce texte, merci. Le président Alizard. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je me réjouis que cette proposition de loi de notre collègue, Samantha Cazebonne nous a permis de débattre dans cet hémicycle de la stratégie du gouvernement visant à doubler les effectifs de l'enseignement français à l'étranger à l'horizon 2030, le Sénat soutient cet objectif ambitieux pour les raisons rappelé dans le débat, notamment par notre rapporteur Bruno Sido intéressant environ 3 millions de Français expatriés, le réseau d'enseignement français à l'étranger par ailleurs l'un des instruments les plus plus efficaces dont du disposons en termes d'influence pour préserver mais aussi développer le rayonnement de la langue et de la culture française sur tous les continents, alors que cette influence est très contesté, notamment sur le continent africain, lutter contre la désinformation nécessite de faire oeuvre de pédagogie, d'expliquer notre vision du monde de diffuser notre narratif, comme le font de façon très décomplexée des pays comme la Russie, la Chine, mais aussi les États-Unis ou le Royaume-Uni, l'Europe et je crois dans ce domaine beaucoup trop discrète, c'est pourquoi la Commission a souhaité mettre l'accent dans ce débat sur la francophonie nos outils de diplomatie culturelle ne doivent pas perdre de vue quelques évidences nous n'accepterons aucun recul face à l'envahissement de la langue anglaise, pourquoi le anglais est-il toujours autant utilisés dans l'Union européenne, malgré le Brexit l'existence de ce faux espéranto mondial qui est l'anglais, est un facteur d'appauvrissement de la réflexion, nous ne devons donc pas céder sur cette question, la commission je crois par ailleurs améliorer le texte sur la notion de représentativité des fédérations de parents d'élèves sur la priorité à donner à la formation des personnels ou encore sur la participation au conseil d'administration de l'AEF de l'association nationale des écoles françaises à l'étranger, mais nous pouvons dire aussi que le Parlement est empêchée d'agir par les règles constitutionnelles de recevabilité sur la question essentielle des moyens financiers de l'EFE et de l'accès à l'endettement, monsieur le ministre, il est urgent, je crois, d'avancer sur cette question et nous attendons des mesures claires pour sortir du bricolage financier actuellement à l'oeuvre avec l'Agence France Trésor, mais aussi des mesures réalistes dans le respect des familles qui, et ça a été régulièrement rappelée sur tous les bancs, p 80 % du coût de fonctionnement de l'enseignement français à l'étranger, je voudrais en conclusion remercié tous les participants à ce débat sous l'autorité bienveillante du président Karoutchi des quelques points de divergence, au-delà des quelques points de divergence, ce texte nous permet je crois, de nous retrouver assez largement sur l'essentiel reste au-delà des grands principes, la traduction dans les faits, c'est comme toujours le travail parlementaire de suivi de l'application des lois qui est pardon une spécialité du Sénat et ce travail devra être mené avec attention, soyez convaincus que notre commission s'y emploiera je vous remercie. J'ai eu un moment d'inquiétude, je croyais que vous aviez encore une feuille, monsieur le président, très bien, non, mais comme il y a un autre texte, derrière c'est pas que je voulais vous précipiter mais il y a un autre texte derrière donc. Allez, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe RDPI sur l'ensemble du texte, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Résultat du scrutin sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence Nombre de votants : 342 Nombre de suffrages exprimés 330 pour l'adoption 330 contre 0, le Sénat a adopté. Merci à chacun, merci monsieur le Ministre et changement d'équipe, nous reprenons la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée visant à combattre le harcèlement scolaire. Madame la ministre bonjour dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 3 ter, l'article 3 ter supprimés après l'article 3 ter l'amendement 16 Madame bourra. Allez-y. Les assistants d'éducation sont des piliers indispensables au maintien du climat scolaire sera présent en dehors des cours au pause méridienne récréation pendant les intercours, ils sont dotés d'une vision complète de la relation inter-élèves et perçoivent plus rapidement les prémices du harcèlement, permettant ainsi d'en limiter l'installation dans la durée, toutefois le droit en vigueur les contraint à quitter l'établissement dans lequel ils exercent au-delà d'un délai de 6 ans maximum cette précarité ne correspond souvent pas aux besoins des chefs d'établissement, désireux de s'appuyer sur des professionnels qui connaissent les réalités de leur environnement, ni aux caractéristiques du harcèlement scolaire celui-ci appelle une alerte immédiate dès lors que le phénomène s'installe et une connaissance longue de l'environnement scolaire, cela paraît d'autant plus décalé que les AED ne sont plus de simples surveillants et que la création de leur corps en 2003 procédé déjà d'une volonté d'adaptation aux réalités nouvelles du second degré, cet amendement vise donc à permettre au personnel AUD ayant exercé pendant 6 ans en cette qualité de poursuivent leur mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cet assouplissement du droit existant doit ainsi permettre au chef d'établissement, de pouvoir continuer à bénéficier d'une ressource humaine précieuse. Merci monsieur le président, madame la ministre, bienvenue, alors on a beaucoup parlé ce matin, des élèves, un petit peu des parents beaucoup des enseignants, on a parlé des chefs d'établissement, on a parlé de médecine scolaire et de santé scolaire Monsieur l'on pratiquement pas évoqué le cas des assistants d'éducation, or, comme le dit très bien Madame ils ont un rôle clé dans la lutte contre le harcèlement scolaire parce qu'ils sont particulièrement proches et le fait de vouloir effectivement leur permettent d'avoir une mission plus longue, s'ils le souhaitent eux-même, c'est une excellente chose, donc la Commission à l'unanimité, déclare que cet amendement aura un avis très favorable. Bon avis favorable, ça m'aurait convenu très bien voilà madame la ministre, si vous avez le même avis, autant le dire tout de suite. Exactement, monsieur le président, c'est un avis de sagesse. Merci, allez sur l'amendement 16 avis favorable de la commission sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté. à l'article 4 2 2 amendements de rédaction globale de l'Arctique, j'imagine le 38 Madame avait. Alors Monsieur le Président, cet amendement tend à réintégrer la reconnaissance du harcèlement scolaire et universitaire comme un délit autonome parce que le harcèlement scolaire ne bénéficient pas, dans ce cas du même interdit symbolique que le harcèlement au travail, sanctionné, quant à lui par un article autonome du code et par de lourdes peines, il paraît nécessaire de poser un interdit clair et cohérent, via un article autonome et c'est ce travail que nous avons également fait récemment concernant les thérapies de conversion cette spécificité permettra aussi une meilleure identification du fameux phénomène la circonstance aggravante n'est pas adapté à l'essence spécifique du harcèlement scolaire en ce qu'elle semble ignorer ses spécificités, en effet, le harcèlement scolaire toc, tout comme le harcèlement au travail ou le harcèlement au sein du couple font référence à des violences qui surviennent dans un environnement duquel il est difficile pour la victime de s'extraire, je vous remercie.

afin de lui apporter toute la substance nécessaire identifié par les acteurs de terrain que sont les associations, les magistrats et les juges et les policiers et gendarmes, le 7ème alinéa de l'article 222 33 2 2 du code pénal, cliente une circonstance aggravante en cas de harcèlement moral sur mineur de moins de 15 ans n'est pas appliquée dans la réalité des faits puisque cette circonstance aggravante repose sur une définition du harcèlement moral, dit entrant d'adulte qui ne prend en considération ni la diversité des typologies de harcèlement, ni la dynamique de groupe, propre au harcèlement scolaire recréer une circonstance aggravante n'aurait donc que peu de sens dans l'utilité même du traitement juridique des faits de harcèlement scolaire il conserverait ainsi le statu quo actuel, pour rappel, bien qu'il est nécessaire d'assortir ce délit d'une peine financière pourra sortir un quorum de peine, celui-ci étant applicable par la justice des mineurs, il ne sera pas envisager une telle condamnation mais bel et bien la prononciation d'un dispositif réparatrice et constructive pour l'enfant, auteur des faits, le suivi de soins thérapeutiques ou encore le suivi d'un stage de sensibilisation et responsabilisation au harcèlement scolaire, c'est le sens d'ailleurs de l'un de mes autres amendements. Malgré l'exclusion et qui sera soumis. Alors les amendements 38 et 31 rectifié se distingue quand même tous les 2 sur un point sur la possibilité de l'un d'inclure ou pas de chance spécifique du harcèlement lié au personnel sur les élèves, donc l'amendement 38 rétabli le texte de l'Assemblée et le 31 dans une Guiness, on distingue sur ce point-là, alors on a déjà eu l'occasion d'avoir longuement ces discussions sur cet article, et comme vous le savez, la commission des lois, est opposé à la création d'un délit spécifique en cohérence, d'ailleurs avec la police, la position de la mission d'information à la cage avait participé avec vous madame le rapporteur qui était là, sur ce sujet, vous étiez pas favorable à un délit spécifique, donc je reprendrai pas les arguments que nous avons développé ce matin et, par ailleurs, le périmètre proposé par cet article pose un certain nombre de problèmes et les 2 amendements proposent de revenir sur le texte de l'Assemblée nationale et de proposer des sanctions assez lourde, sachant que il ne faut pas oublier qu'il y a les victimes et le harceleur et qu'il y a beaucoup à un travail de prévention aussi à mettre en place sur ce sujet, nous pensons que tout cela est trop restrictive par rapport à la réalité des faits de harcèlement ce c'est bien de toucher les élèves et les enseignants, donc il n'est pas souhaitable de de réécrire en tout cas de réinstaller dans ce texte, ce que nous avons supprimé en tout cas c'est notre position, par ailleurs, le quantum de peine proposée de 3 ans à 10 ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende paraît quand même pas pour la commission des lois trop élevé par rapport à l'objectif affiché de la proposition de loi qui est de prévenir parce que c'est important de prévenir le harcèlement scolaire et non de sanctionner par de lourdes peines de prison, les mineurs qui peuvent s'en rendre coupable, je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un travail important, donc il est donc apparu aussi à la commission, conformément à la position de la commission des lois de la culture pendant qu'il est nécessaire aussi de distinguer ce qui relève du harcèlement entre élèves et les faits impliquant des adultes, ça nous y sommes attachés, ce n'est pas le même sujet, ce n'était pas la même prise en charge des choses, ces faits doivent être sans sonner mais ne peuvent être appréhendées en tout cas pour nous de la même manière, donc il ne nous paraît donc pas possible de rétablir le texte de l'Assemblée nationale et donc, nous vous proposons de maintenir ce que nous avons souhaité à la commission des lois, d'avoir une circonstance aggravante dans le droit existant, donc je vous proposerai chers collègues soit le retrait de vos amendements soit des maîtres pour les deux un avis défavorable.

et comme le 2ème amendement le 31 va également dans le même sens, c'est un avis de sagesse, même si le l'amendement de Madame avait juste pourquoi nous avons besoin de cet amendement parce que le harcèlement scolaire et spécifique, il permettra en réalité de quantifier le fléau du harcèlement scolaire qui est très très spécifique qui brisent parfois des jeunes, des adolescents et si nous n'avons pas la la quantification si nous ne pouvons pas évaluer le nombre de jeunes qui sont victimes de ce harcèlement scolaire alors ça restera en réalité trop large et je crois que finalement ce fait social grave qui, aujourd'hui, mais malheureusement au drame n'aura pas suffisamment d'éléments pour lutter et amener les politiques de prévention les plus justes, donc c'est un avis favorable à l'amant 38 et un avis de sagesse, à défaut, la maman 31. Merci, je vais mettre aux voix d'abord. Oui, madame. Excusez-moi, voilà merci Monsieur le Président, je voudrais simplement dire que même si le rapport en effet il n'était pas pour le délit de harcèlement et vous l'avez rapporté Madame

voilà donc retiré pour le mien. Donc le 31 et retiré je mais on voit le 38 qui a un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté.

Article 4 bis, le 18 madame la rapporteure coordination gouvernement favorable mais aux voix l'amendement 18 de la commission avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est con, il est adopté 2 amendements en discussion commune le 21 qui le défend oui. Merci monsieur le président je vous présente l'amendement de notre collègue Pierre-Antoine Levi cet amendement porte sur l'article IV bis qui. Prévoit entre autres que les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l'exige et que celle-ci porte sur un Crime ou sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement, d'une durée égale ou supérieure à 3 ans or pour renforcer l'arsenal législatif contre le harcèlement et le et combattre sous toutes ses formes, il est nécessaire d'aligner cet article IV bis alinéa 17 sur l'article 222 tiré 33 tiré qui prévoit que certains actes ou comportements constitutifs du harcèlement sont punis d'un an d'emprisonnement. Monsieur Lévy propose donc de réécrire l'article 4 bis à il y a 17 pour renforcer les moyens de la justice dans son ensemble à l'encontre de ces faits délictuels de harcèlement. C'est le 51 du gouvernement Madame la ministre. qui a mis réellement en évidence un besoin en tout cas une problématique et donc du coup la le la : le gouvernement propose dans la philosophie de l'amendement et des travaux de la de la de la commission et les travaux du sénateur Lévy hé bien simplement une écriture un peu différente, mais qui permet de fixer un seuil, y a un an lorsqu'il s'agit de réquisition qui ont pour seul but d'identifier l'auteur du délit commis par Internet, nous en avons besoin, nous connaissons le fléau aujourd'hui du cyber-harcèlement et en réalité, c'est pour être opérationnel. la Commission va me donner la vie sur les deux amendements puis le gouvernement sur le 21 oui. Donc moi j'ai effectivement échangé avec notre collègue Me Lévy pour lesquels nous avions effectivement hésité lors de la commission parce que son amendement fragilisé un peu son application par sa rédaction et et nous avions effectivement émis un avis défavorable, parce que voilà, son contenu nous poser quelques difficultés sur son application, alors effectivement on a échangé avec la Chancellerie, échanger avec le cabinet de ce ministre

de l'amendement du gouvernement qui effectivement correspond aux souhaits de monsieur Lévy au sein du gouvernement avec un avis favorable de la commission. vous retirez l'amendement de il est retiré, merci donc, ben il reste que le vôtre, donc par définition, est ce que vous avez le même avis au profit du vôtre. Jusque-là, Madame la Ministre, j'avais conscience le 51 du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre, il est adopté. L'article 4 bis. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Après l'article 4 bis, un amendement 32 Madame bourra. cette lacune est d'autant plus dommageable que le harcèlement scolaire et en particulier le cyber harcèlement s'étendent au collège mais aussi au lycée en 2021 sur les 22 victimes mineures ayant attenté à leurs jours, 8 étaient âgés entre 16 et 18 ans, maintenir une circonstance aggravante pour les seuls mineurs de 15 ans n'apparaît donc pas adaptées aux réalités sociétales nouvelle faisant apparaître une extension du phénomène à toutes les tranches d'âge et donc une nécessité de le stopper Net, quel que soit loi l'âge du mineur concerné, cet amendement vise donc à combler ce vide juridique afin de couvrir l'ensemble du spectre des potentielles victimes mineures. Alors effectivement le droit pénal sanctionne en général plus sévèrement les infractions sur les mineurs de moins de 15 ans qui sont sujets plus vulnérables, donc la question posée par notre collègue aujourd'hui une heure moins importante pour la protection des 15 18 ans, je voulais simplement rappeler qu'en 2018 une circonstance aggravante concernant tous les mineurs témoins de faits, et non seulement les mineurs de 15 ans a été ajoutée à l'article sur le harcèlement, dès lors, effectivement, il nous paraît tout à fait logique détendre la circonstance aggravante concernant les victimes à tous les mineurs, donc c'est un avis favorable de la commission. Merci, il y avait du gouvernement, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, le gouvernement a un avis particulièrement réservé sur cet amendement et à-t-elle plutôt au retrait, mais compte tenu de la vie, je crois, de la commission, ça sera du coup un avis défavorable. Très bien, je mais on voit le 32 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté. à l'article 5 le 19 coordination madame le rapporteur. Coordination. Avis du Gouvernement favorable je mais au voit le 19 de coordination qui est pour. Qui est contre, il est adopté, jamais aux voix, l'article 5 qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Article 6 avec 3 amendements identiques de rétablissement d'abord le 11 qui le défend. Oui, madame. Oui, monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues par cet amendement, nous souhaitons rétablir la possibilité de mise en oeuvre dans le cas des différentes procédures judiciaires pour harcèlement scolaire ou universitaire de stage de responsabilisation, à la vie scolaire, comme le prévoyait la proposition de loi initial, ce dispositif rejoignaient les préoccupations de la mission d'information sénatoriale qui suggérait le développement des stages de la PJJ, pour les personnes condamnées et le développement des travaux d'intérêt général, traitant spécifiquement du harcèlement pour les auteurs de harcèlement, de façon générale, la mission d'information avait estimé que la prévention était préférable à la sanction dans les affaires de harcèlement, les stages de citoyenneté ou de formation civique avec des mentions spéciales de sensibilisation lié au risque de harcèlement scolaire ordonnée, soit par le procureur de la République, soit par la rigidité sur pénale ne constitue certes pas des mesures préventives mais apporte quand même une réponse d'ordre pédagogique aux délits de harcèlement à mes yeux préférable à des sanctions lourdes l'accomplissement d'un texte stage permet aux jeunes de mieux prendre conscience de ses actes de le responsabiliser, voire même de lui permettent de reprendre confiance et de re-acquérir un peu d'estime de soi, grâce aux missions réalisées durant ce stage, je vous remercie. Merci. Le 30 identique Madame. Oui en Oui en effet il est identique, mais là franchement, je pense que c'est important de créer un stage de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ce qui s'inscrit dans une démarche de prévention, comme l'a dit ma ma collègue, ce dispositif est primordiale car participe à la reconstruction psychologique des enfants harcelés et de leur famille le présent amendement envisage donc un dispositif avisé réparatrice et constructive pour l'enfant, auteur des faits, le suivi d'un stage de sensibilisation et les sensibilisation au harcèlement scolaire ne sont importants, merci. Merci le 39 identique Madame avait. Mes collègues ayant très bien argumenté, il est défendu. Merci et la commission sur les trois identique. Alors la commission effectivement n'est évidemment pas hostile à des stages et des des peines qui peuvent effectivement donner un peu de sens à ce qui est à ce qui est proposé, sauf que la commission des lois, elle est attachée extrêmement attaché à bien faire la différence entre ces 2 heures de la loi et de l'or du règlement, or, or tout ce qui nous a été présenté là qui est important, qui a du sens, est du domaine du règlement, c'est pour ça que la commission effectivement s'est positionné avec la suppression de ce qui est proposé dans le texte de loi qui est de l'ordre réglementaire, on essaye de pas surcharger les lois par du règlement, donc c'est pour ça que nous avez j'ai on propose un avis défavorable sur ces trois amendements.

que nous n'aurions pas apprendre et finalement des vies qui ne serait pas brisée, c'est pour ça que le gouvernement est favorable, parce qu'il est, il lui paraît opportun d'inscrire dans la partie législative du code de la justice pénale des mineurs que les stages pouvant être prononcée contre ce qui serait finalement qui aurait commis des de 6 infractions scolaire est une à mon avis, à une vraie avancée dans cette lutte contre le harcèlement et le cyber harcèlement. Merci, je vais mettre aux voix, ces trois amendements identiques avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement. Qui est pour. Merci qui est contre. Ils sont rejetés. Je mais on voit l'article 6 qui est pour. Qui est contre, il est adopté. L'article 7 été supprimée mais j'ai un amendement et 3 sous-amendements de rétablissement donc le 12 Madame Voynet. Monsieur le président, par cet amendement, nous souhaitons, d'une part rétablir le dispositif de l'article 7 issu des travaux de l'Assemblée nationale, mais également aller plus loin et le compléter, il est urgent que les fournisseurs d'accès Internet et les hébergeurs de services soient davantage responsabilisés face au fléau du cyber harcèlement qui se propage et se démultiplie sur les réseaux, l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique porte déjà obligation aux fournisseurs d'accès, hébergeur de services de communication au public en ligne de lutter contre la diffusion de certains contenus favorisant différents crimes et délits, tels l'apologie, la négation la banalisation des crimes contre l'humanité, la provocation à la la commission d'actes de terrorisme et leur apologie, l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard des personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap, ainsi que de la pornographie enfantine, l'incitation à la violence sexuelle ou sexiste, les atteintes à la dignité humaine, il me semble donc tout à fait logique d'inclure le harcèlement scolaire et universitaire dans la liste des contenus contre la diffusion desquels ces prestataires devront lutter, par ailleurs, nous souhaitons aller plus loin que cette simple obligation assez vague de lutte ainsi, outre le rétablissement de l'article voté par l'Assemblée, nous proposons de compléter le dispositif des obligations des prestataires de service du Net en reprenant une proposition de la mission d'information, il s'agit d'obliger ses prestataires à présenter périodiquement à leurs utilisateurs de courtes vidéos de sensibilisation sur les bons usages du numérique, la prévention du cyber harcèlement et les moyens pour les victimes de réagir, la mission d'information avait en août souhaité aussi renforcer l'accessibilité des sites de sensibilisation au harcèlement et d'accompagnement des victimes et ces dispositions sont davantage de nature réglementaire que législatives, je suis heureuse de constater que ma collègue Céline voulez respect rogner partagent mes préoccupations ces sous-amendements qui visent notamment à prévoir une régularité dans la diffusion par les dix prestataires de ces vidéos à prévenir les usagers des peines encourues en cas de mauvais usage des réseaux répondent à des préoccupations partagées, j'espère que le Sénat dans sa majorité votera cet amendement et ses sous-amendements, je vous remercie. présenter déjà les sous-amendements de Madame vous l'esprit renié mais je pense qu'elle va vouloir quand même le présenter elle-même les 3. Non, non, mais vous pouvez même prendra micro Madame Boulay-Espéronnier je dis ça, moi vous savez. Si Monsieur le Président, donc le 1er défendu et les 2 autres j'allais présente donc dans la foulée, hein, c'est ça, donc le 2ème complètent le dispositif proposé à l'article 7 en demandant aux réseaux sociaux de sensibiliser leurs usagers sur les peines encourues en cas de cyber-harcèlement afin d'attirer leur attention sur les conséquences que peuvent avoir un mauvais usage de ces plateformes et l'amendement 46 rectifié dit que, aujourd'hui, les conditions d'utilisation des réseaux sociaux sont illisibles, tant pour les enfants que pour les parents ce sous-amendement propose donc d'obliger les prestataires de services de communication en ligne de présenter de manière explicite les extraits de leurs conditions générales d'utilisation relatives au harcèlement afin de sensibiliser leurs utilisateurs au bon usage de ces plateformes. Merci, cher collègue, avides de la rapporteure sur l'amendement et 3 sous-amendements. Alors, sur ces sujets effectivement du cyber-harcèlement et et et le monde peut-être certains d'ailleurs d'efficacité des plateformes, je crois qu'on partage tous l'inquiétude que vous nous avez exposé chers collègues et et et que notre collègue, a posé aujourd'hui nous avons souvent eu ces discussions lors du la discussion de la loi via lors de la discussion principes de la République parce que nous, nous avons fait ensemble le gouvernement le Sénat fait avancer déjà les choses mais il faut, oublier que c'est pas la France, dans son petit coin tout seul qui va régler ça et nous pensons qu'effectivement, et nous l'avons souvent dit ici la réponse réside dans un cadre européen, qui est d'accord en cours d'élaboration, aujourd'hui, entre autres, avec des mesures sur lequel les pays, les pays européens réfléchissent donc c'est pour ça que nous avons, moi je vais vous proposer soit de retirer vos amendements soit dit donner des avis défavorables, parce que ce sujet là un sujet important doit être pris en charge par l'Europe, parce que c'est l'Europe qui doit trouver effectivement des réponses sur ces sujets, la France tout seule ne pourra pas les régler malheureusement. Madame la Ministre. Monsieur le président, il se trouve que, aujourd'hui, le sujet du cyber harcèlement en particulier, c'est ce qui ne permet plus de répit aux jeunes qui se qui subissent un harcèlement scolaire et cette frontière est tellement tenu que par l'usure, malheureusement les drames arrivent le gouvernement en réalité comprend totalement l'argumentation posées par la rapporteure et effectivement ça appellerait à à la assure mais dans le fond, ça sera un avis de sagesse pour l'ensemble des amendements parce que je crois qu'il faut effectivement montré cette envie de ne se priver d'aucun moyen pour lutter contre le harcèlement et le cyber-harcèlement en particulier. Bien. Madame Mellow. Merci monsieur le président, oui, je voudrais insister sur le fait que de nos jours, il n'y a pas de harcèlement sans cyber harcèlement c'est extrêmement grave, parce que comme Madame la ministre vient de le dire, il y a un continuum entre le ce qui se passe dans l'établissement scolaire et la sphère privée, donc, même si nous savons que les plateformes et les hébergeurs ne sont pas domiciliés dans notre pays et qu'il y a des travaux qui ont été commencés par l'Europe pour pouvoir y remédier, il faut quand même insister quand même insister sur ce point et faire figurer dans notre loi la la nécessité que les hébergeurs et les fournisseurs d'accès interviennent lorsqu'il y a du harcèlement. Merci madame Boulay-Espéronnier. Si oui, étant donné qu'il y a un consensus dans l'hémicycle sur ces sujets, j'aimerais vraiment que ces amendements soient votés parce que l'idée, c'était vraiment de mettre les plateformes et les hébergeurs, les éditeurs devant leurs responsabilités, souvent elles en sont exempts, cette histoire du cyber harcèlement, elle est fondamentale est au coeur du problème parce qu'il y a des multiplie par 50 ou par 100, les problèmes de harcèlement, on le sait et on sait aussi qu'il ne faut pas faire preuve d'angélisme, puisqu'on sait que c'est les modèles économiques des plateformes qui sont en cause et c'est donc très, très important à mon sens d'inscrire dans le texte là aujourd'hui que leurs responsabilités vraiment au coeur du problème. Je vous remercie, merci, je vais donc mettre aux voix successivement madame Vaneck pardon. Monsieur le président je je réponds à Madame la rapporteure, bien sûr que nous attendons une prise en compte de l'Europe. Mais nous avons le devoir d'imposer, nous en France aux plateformes de prendre en compte cette cette question et d'agir. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fond, mais les outils, à nous petits français dans notre coin, ça, c'est pas comme ça, malheureusement, qu'on va le gérer, on peut écrire dans la loi qu'on a des intentions, je pense que la prise en compte réelle des contraintes des contraintes au niveau de l'Europe, il y a que ça comme solution voilà parce que on peut effectivement écrire qu'on souhaite qu'il prenne conscience bah oui vont vous écrire qui vont prendre conscience, mais s'il y a pas des contraintes fortes européennes qui puisse les sanctionner, tout ça c'est du domaine du souhait mais ça ne suffira pas, vraiment, il faut qu'on en soit conscient, on a souvent eu cette discussion aussi, il faut en avoir conscience que le fait qu'on est qu'on en discute aujourd'hui c'est important, mais au niveau européen, il va falloir que ça bouge beaucoup plus, parce que les plateformes de toute façon, elles ne sont pas ici ne sont pas chez nous, comment on va imposer à l'Irlande, un certain nombre de choses si l'Europe n'a pas de règles, voilà par exemple. Bien, alors je vais mettre aux voix maintenant successivement les sous-amendements puis l'amendement, je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable que l'avis du Gouvernement c'est sagesse c'est ça Madame la Ministre, alors d'abord le 46. Qui est pour. Oui, j'allais dire, madame vous l'espériez, c'est le vôtre. qui est contre. Qui est contre. Il est adopté le. 45 même chose donc défavorable de la commission sagesse du gouvernement qui est pour. Merci qui est contre. Il est adopté. Le 44 E même chose donc avis défavorable de la commission sagesse du gouvernement qui est pour. Il est adapté, Il est adapté, et enfin l'amendement. 12 ainsi sous-amendé, si je puis dire, avec un avis défavorable de la commission sagesse du gouvernement qui est pour. Merci qui est contre. Adopté, l'article 7 est ainsi rédigé est rétabli après l'article 7 le 22, oui, je vous en prie. et leur effet amplificateur du harcèlement, mais il faut aussi penser aux nombreuses applications et messagerie aujourd'hui qui laissent les jeunes victimes de harcèlement, quasiment sans répit, alors il y a des dispositifs qui existent d'ores et déjà, mais il nous semble nécessaire de les renforcer, c'est le sens de cet amendement pour protéger mieux encore nos jeunes merci. Alors c'est vrai qu'chers collègues, on en a discuté ensemble et et on comprend la motivation de votre amendement qui souhaite que les outils de lutte soient clairement exposés ça on entend, on entend bien, c'est que il semble cependant que cela soit déjà satisfait en droit, c'est la mise en oeuvre effectivement de tous ces procédés de tous ces objectifs, hein, et de ces outils qui pêche et qui repéré répéter l'obligation, parce que cela, c'est l'objet de cet amendement, c'est de rappeler les obligations ne changera malheureusement pas grand chose à la situation actuelle, donc, et ce qui nous semble important, c'est que les pouvoirs publics doivent mener un travail plus étroit avec les plateformes parce qu'aujourd'hui il y a que ça qui peut être efficace pour parvenir à mieux protéger ça, on est conscient ça, c'est une nécessité de le rappeler, de le redire, mais que ce n'est pas du domaine effectivement du contexte de la loi de l'écrire ainsi, et donc je vous proposerai chers collègues soit le retrait de votre amendement soit d'émettre un avis défavorable. Madame la Ministre, ma vie.

Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, y a-t-il des demandes d'explications de vote, madame anez. Monsieur le président, mes chers collègues, Madame la ministre, le texte de la PPA le à l'issue de son examen par les 2 chambres leur permettent de davantage appréhender et punir les phénomènes de harcèlement scolaire grâce à un traitement Haddock et des peines, il permettra également d'effectuer davantage de sensibilisation en direction des élèves et de tous les acteurs de la communauté éducative et de formation des personnels concernés, de nombreuses propositions de la mission d'information sénatoriale ne trouve aucune concrétisation dans ce texte, la plupart étant de nature infra-législatives il reviendrait donc on gouvernement au gouvernement, pardon, de prendre rapidement les mesures réglementaires nécessaires à leur application, nous ne pouvons pas nous opposer au texte issu des travaux parlementaires, mais s'il faut bien constater que les les débats au Sénat ont plutôt abîmé le texte notamment par l'adjonction de dispositions concernant l'instruction en famille le phénomène très graves de harcèlement pouvant servir de prétexte pour renforcer ce monde ce mode d'instruction que nous considérons comme inégalitaire, le harcèlement scolaire n'est même pas identifiés comme tels mais comme menace à l'intégrité physique et morale, notion beaucoup plus large et flou que le harcèlement nous saluons la refonte de l'article 4 qui correspond davantage aux orientations de la mission d'information et déplorons que 3 des 4 amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain n'ait pas été repris repris par le Sénat, alors qu'ils avaient pour objet de mieux contrer le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement pour autant la gravité du problème qui peut toucher tous nos enfants et la nécessité d'avancer pour mettre un vrai terme à ce fléau, nous amène à voter en faveur de ce texte, je vous remercie. Merci monsieur le président, nous arrivons donc à l'issue de l'examen des articles de cette proposition de loi nous partout sont tous sincèrement le même dessin éradiquer ce fléau que constitue le harcèlement scolaire cependant force est de constater que nous ne sommes pas d'accord sur la nature des dispositifs qui nous permettront d'atteindre cet objectif commun : notre groupe considère qu'il est indispensable d'inclure les adultes dans le Champ du harcèlement scolaire que la création d'un délit autonome du harcèlement scolaire est nécessaire et nous croyons aussi au stage de la responsabilité de la à la vie scolaire par conséquent au regard des modifications importantes notre groupe s'abstiendra sur ce texte en l'état, je vous remercie. Merci monsieur le président, les travaux de l'Assemblée nationale qui ont donné lieu à une PPL 100 complémentaires à ce qui a mené la mission d'information sénatoriale, je crois qu'il est, il est important d'attirer l'attention sur le harcèlement qui est un fait de société extrêmement grave et tout, toutes les mesures que nous avons listé dans le dans le le rapport suite à la mission que nous avons menée en 2021 devraient être petit à petit appliqué car je le rappelle encore en présence de Madame la ministre, ce sont des mesures pragmatiques, qui ne nécessitent pas vraiment des moyens importants, c'est simplement une question de volonté pour les mettre en en oeuvre, il s'agit de prévention essentiellement parce que vraiment, la prévention est le maître-mot pour lutter contre le harcèlement scolaire ensuite, bon, il y a la détection, évidemment, et ça, ça dépend de la formation et le traitement à la fois des des victimes et des auteurs, je rappelle que l'école prépare les citoyens de demain il est inadmissible qu'il y a autant de faits de harcèlement dans les établissements scolaires, j'espère que les les nos collègues députés prendront en compte toutes nos remarques, en particulier en ce qui concerne le cyber harcèlement qui est extrêmement important de nos jours, je vous remercie. que que nous voudrions soutenir ce cette PPL parce que tout ce qui ira vers une reconnaissance et une pénalisation du du harcèlement doit l'être, alors, on regrette vraiment qu'on ne poursuit pas tous les harceleurs les adultes comme comme les autres élèves, je pense que c'était quelque chose d'important malgré tout, on espère que les choses s'amélioreront et tout ce qui va dans le bon sens est un petit pas à gagner l'autre chose aussi bon qu'on parle absolument de cyber harcèlement c'est tout le harcèlement que nous condamnons et le cyber harcèlement étant harcèlement, donc on n'en faisait pas une vraiment un sujet de de rupture donc je, on espère que les mentalités évolueront que les avis aussi progresseront et qu'on pourra vraiment condamner progressivement tous les harceleurs adulte comme scolaire. Merci madame la présidente Billon. Merci monsieur le président, le groupe Union centriste votera cette proposition de loi amendée par le Sénat, je remercie sincèrement les rapporteurs Jacqueline Eustache-Brinio et Olivier Paccaud pour leur travail sur ce texte, moi je voudrais dire que la nouvelle disposition proposée consacrant à harceler harcèlement entre pairs cette c'est une bonne chose, une définition trop large du harcèlement scolaire incluant notamment les personnels de l'Éducation nationale aurait forcément amené des dérives donc ce texte est un signal fort qui est envoyé aux victimes l'harcelé, je pense aussi aux victimes, bien entendu, mais à leur famille, ce soir, c'est un signal fort, mais ce n'est qu'un 1er pas car ce fléau est un phénomène d'une grande ampleur qu'on ne mesure probablement pas encore complètement le Sénat a intégré le cyber harcèlement ce cyber harcèlement qui ne laissent aucun répit aux victimes, lutter contre le cyber harcèlement, vous l'avez dit madame la rapporteure ne se fera qu'à qu'à grande échelle, on ne pourra pas le faire seul, lutter contre le harcèlement sera effectif aussi quand on accordera des moyens à la médecine scolaire pour détecter, informer, alerter et accompagner les victimes, lutter contre le harcèlement scolaire c'est assurer la formation de tous les acteurs qui sont au contact des enfants, donc la question des réseaux départ la de forme reste entière est cruciale, nous avons encore du travail, madame la Ministre Mesdames et messieurs, chers collègues, sur ce sujet, merci. Merci madame brûle, Merci monsieur le président, je confirme que notre groupe votera ce texte tels que retravailler ici par le Sénat et je voudrais à mon tour saluer la qualité du travail de nos rapporteurs, en particulier sur l'article IV qui était celui qui, pour nous faisait le plus de problèmes dans sa version originale parce que portant des peines disproportionnées mal ficelée, si je peux l'écrire les dire en ces termes, il aurait été de fait inopérants, or chacun et je crois qu'on a témoigné tout cela volonté aujourd'hui a envie de lutter de manière efficace contre le harcèlement scolaire je ne souhaite pas que ce qui reste ce soir de notre débat, ce soit l'idée les les personnels de l'Éducation nationale soit épargné parce que le délit de harcèlement moral existe et qu'il peut être mobilisés dans les cas rares, fort heureusement, mais qui existe de harcèlement d'adulte envers les enfants et puis je mets une amicale pression sur nos rapporteurs pour la CNP, parce que je crois que ce texte est désormais très équilibré, très opérants, j'y reviens, il ne s'agit pas juste de faire de l'affichage, il s'agit de se donner des moyens efficaces de lutter contre le harcèlement scolaire il y a des lignes rouges, je ne vais pas les énumérer : pour nous, mais je suis convaincu que vous aurez à coeur de défendre la position qui est a été celle du Sénat et je vous en remercie. Merci, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans La Commission a rédigé ainsi l'intitulé : proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyber Hassan. Qui est contre. Qui s'abstient. La proposition de loi est adopté. Mes chers collègues, annonces paroissiales, ça n'avait pas un moment non, non, mais si vous voulez partir d'hésiter pas. Par lettre en date de ce jour, le gouvernement qui n'hésite pas, demande le retrait de l'ordre du jour du mardi 8 février du projet de loi étendant et adopta la fonction publique des communes de Polynésie française. Certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et son remplacement par l'examen des conclusions de la CMP sur le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante initialement inscrite à l'ordre du jour du 16 février par ailleurs le même gouvernement demande l'inscription à l'heure du jour du mardi 15 ans 1er Point de l'Ordre du jour de l'après-midi de quatre conventions internationales relatives à l'approbation de l'accord entre la République française et l'État du Qatar, établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du monde de foot de 2022 autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, autorisant l'approbation de l'accord entre la République française et la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, autorisant l'approbation de l'accord entre la République française et l'État du Qatar relatif au statut de leurs forces, demande également à l'inscription à l'Ordre du jour du jeudi 17 de la 2ème lecture du projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi du 2 août 2019 relatives aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace, l'examen des conclusions des CMP ou la nouvelle lecture des propositions de loi visant à combattre, justement, le harcèlement scolaire pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur et l'examen des conclusions de la CMP sur la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône ainsi que la proposition de loi visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales acte et donner de ces demandes pour l'examen de ces textes nous pourrions prévoir de siéger le jeudi 17 février à 10 heures 30, 14 heures 30 éventuellement le soir à la demande du gouvernement, qui décidément n'hésitent plus, nous pourrions examiner les quatres conventions internationales selon la procédure simplifiée, le délai limite pour la demande de retour à la procédure normale s'est fixé au vendredi 11 février à 15 heures pour l'examen du projet de loi relatif à la collectivité européenne d'Alsace nous pourrions fixer le délai limite du dépôt des amendements de séances au lundi 14 février à 12 heures nous pourrions également prévoit une discussion générale de 45 minutes en cas de nouvelle lecture sur la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire nous pourrions prévoit un délai limite pour le dépôt des amendements séance au lundi 14 février à 12 heures ainsi qu'une discussion générale de 45 minutes pour l'examen de la proposition de loi visant à simplifier les experts forestiers aux données cadastrales nous pourrions fixer le délai limite du dépôt des amendements de séance au lundi 14. Février à 12 heures, y a-t-il des observations, c'est une demande. Oui enfin récurrente mais bon oui j'imaginais, il en est ainsi décidé, mes chers collègues, je vais lever la séance en remerciant Madame la ministre madame et monsieur le rapporteur et l'ensemble des collègues qui sont restés prochaine séance mardi 1er février à 14 heures 30 pour le débat sur les menaces que les théories du wokisme font peser sur l'université, l'enseignement supérieur et les libertés académiques, la séance est levée.